L'ordre du jour appelle une déclaration du gouvernement, suivie d'un débat en application de l'article 50 la Constitution sur la politique énergétique et nous aurons donc la séance et je vais donner immédiatement la parole à Madame la première ministre Élisabeth Borne.

Merci monsieur le président, Mesdames et messieurs les sénateurs. L'énergie est au coeur de notre quotidien. Chaque transition énergétique a apporté des changements majeurs dans nos sociétés. Nous sommes en train de vivre une de ces transitions. Et nous devons la mener avec détermination et rapidité. Nous devons l'amener avec justice et de manière, en faire une opportunité pour nos vies pour notre économie, pour notre planète. Cette transition est impérative. Dès 2018, le président de la République a chargé RTE d'étudier les différents scénarios devant nous. Et en février dernier à Belfort, il a présenté une stratégie énergétique pour notre pays. Quelques jours plus tard, le 24 février la Russie a envahi l'Ukraine. Par cette décision. Vladimir Poutine a violé les règles internationales agressé un État souverain et déclaré la guerre à nos valeurs. Depuis, le Kremlin a montré qu'il était prêt à tout pour gagner cette guerre. Toutes les exactions toutes les menaces tous les chantages. Et parmi eux se trouvent les exportations de gaz. L'arrêt quasi-total des livraisons de gaz russe vers l'Europe, augmentent les risques de pénurie et provoque une explosion des prix de l'énergie. à cette situation s'ajoutent d'autres tensions. Je pense au pétrole, conséquence de la guerre en Ukraine et du refus des pays de l'OPEP d'augmenter la production. Je pense également Automne aux tensions sur notre production d'électricité. Avec l'arrêt pour maintenance, d'une part de notre parc nucléaire, j'y reviendrai. Bien sûr, ce sont des effets conjoncturels. Mais d'autres s'installe dans la durée. La sécheresse effet du dérèglement climatique, par exemple via limiter notre production d'hydroélectricité. Ce contexte nous impose d'aller plus vite et plus loin. Nous devons accélérer notre transition énergétique, nous devons sortir des énergies fossiles conquérir notre indépendance énergétique et décarboner nos modes de vie et notre économie. Nous devons tous nous mobiliser, c'est notre responsabilité collective. Mesdames et messieurs les sénateurs, face à cette situation critique. Notre 1er devoir est de répondre à l'urgence et de protéger des Français. Notre 1er défi et de faire en sorte que nous puissions traverser l'hiver sans difficulté dès cet été, nous avons pris des mesures pour sécuriser nos approvisionnements, nous avons décidé de porter nos stocks de gaz à 100 Cet objectif est aujourd'hui atteint. Nous avons diversifié nos approvisionnements en nous tournant notamment vers la Norvège, l'Algérie et les États-Unis. Nous avons augmenté les capacités de nos terminaux méthaniers et avec le Parlement, nous avons lever les verrous pour installer rapidement un nouveau terminal méthanier au Havre. Les travaux sont en cours. Ces mesures ont porté leurs fruits et nous sommes aujourd'hui l'une des principales portes d'entrée du gaz en Europe. Cela donne corps à la solidarité européenne. Nous allons être en capacité d'exporter du gaz, notamment vers l'Allemagne tout au long de l'hiver et nos voisins nous livrerons en retour l'électricité dont nous aurons besoin. Dans le même temps, notre parc nucléaire et dans une situation d'indisponibilité exceptionnelle mais conjoncturel. Elle s'explique d'une part par le rattrapage d'une partie des maintenance qui aurait dû se dérouler pendant l'épidémie de Covid. Et d'autre part par un problème dit de corrosion sous contrainte détecté en octobre 2021 qui a entraîné l'arrêt de 12 réacteurs pour contrôle et réparation. Le calendrier de réparation prévoit un redémarrage de ses réacteurs entre aujourd'hui et février je sais, les équipes de tête d'EDF extrêmement mobilisés, et je leur fais confiance pour respecter ce calendrier. Grâce à notre action, grâce à la solidarité européenne et grâce à la sobriété, j'y reviendrai, nous pouvons éviter les pénuries. Dans le même temps, nous devons répondre à une autre urgence et protéger les Français face à l'explosion des factures d'énergie. En Allemagne, en Italie, en Belgique, au Royaume-Uni, les montants payés par les consommateurs ont explosé et les prix ont parfois été multipliés par plus de deux. De notre côté, très tôt, nous avons agi, nous avons mis en place le bouclier tarifaire qui a bloqué les prix du gaz et limiter la hausse des prix de l'électricité. Et. Ce bouclier, nous avons décidé de le prolonger. Grâce à lui, la hausse des factures des ménages sera limitée à 15 % il en est de même pour les factures d'électricité, des très petites entreprises et des plus petites communes. Sans bouclier les prix aurait doublé. Pour nos compatriotes qui se chauffent au fioul ou au bois des soutiens spécifiques ont été décidées. Ces mesures sont les plus protectrices d'Europe. nous les avons complétés d'un chèque énergie exceptionnel pour les 40 % de Français les plus modestes qui sont les plus touchés par la hausse des prix de l'énergie mais protéger, cela ne se limite pas seulement aux ménages. Je connais la préoccupation particulière du Sénat pour les collectivités. Je crois que. Je sais aussi votre attachement à notre vitalité économique et votre inquiétude pour les factures d'énergie des entreprises. Ces préoccupations, ce sont aussi les miennes et celle de mon gouvernement. Ces derniers jours, nous avons pris plusieurs mesures en demandant l'engagement et la transparence des fournisseurs d'énergie. Nous voulons d'abord garantir qu'il n'y ait plus d'entreprises ou de collectivités, son fournisseur. Nous voulons d'autre part, faire en sorte que chacun puisse vérifier qu'on ne lui propose pas d'offres abusive grâce à des indicateurs de prix qui seront publiés par la Commission de régulation de l'énergie. Pour les entreprises, nous travaillons avec nos partenaires européens et la Commission à améliorer les aides mises en place après l'agression russe, à destination des entreprises les plus consommatrices. Quant aux collectivités, qui connaissent des difficultés, les plus fortes, un filet de sécurité a été adopté par le Parlement pour 2022, sa mise en place sera rapide et des acomptes seront versés d'ici la fin de l'année. Comme je l'ai dit, devant vous, la semaine dernière, je souhaite que ce filet de sécurité soit prolongé en 2023 et qu'qui puisse bénéficier à toutes les collectivités. Nous travaillons actuellement à ses contours précis et nous pourrons le présenter rapidement. J'ajoute que face à cette situation difficile, j'ai pris la décision avec le ministre en charge de la cohésion des territoires de porter l'augmentation de la DGF à 320 millions d'euros au lieu de 210 millions d'euros prévus initialement. 7 E au, la première en 13 ans permettra à 95 % des communes de voir leur DGF se maintenir ou augmenter. Et je le dis clairement : aucune collectivité aucune entreprise ne sera laissé dans l'impasse. Mais au-delà de ces mesures, nous sommes au front pour faire baisser les prix de l'énergie. Alors, soyons lucides, les prix du gaz et de l'électricité ne reviendront pas au niveau bas de la période Covid. Mais leur niveau actuel ne sont pas raisonnables, ils sont très excessif par rapport au coût de production et sont tirés vers le haut par des craintes exagérées de pénurie et par la spéculation. Nous voulons ramener les prix à la raison. Nous y travaillons d'abord en européen, l'Europe a déjà agi une obligation de remplissage des stocks de gaz à 80 % a été approuvé, nous sommes déjà à 90 pour 100 au niveau européen et des règles de solidarité entre États membres ont été décidées en cas de pénurie de gaz. Par ailleurs, le conseil des ministres de l'énergie a adopté un règlement qui autorise chaque État membre, à mettre en place une contribution exceptionnelle de solidarité des des entreprises du secteur fossiles et une taxation des bénéfices exceptionnels des producteurs d'électricité. Tout cela va dans le bon sens mais ne suffit pas. Car il faut aussi agir directement sur les prix. Le président de la République est pleinement mobilisé sur le sujet, il s'est entretenu avec la présidente de la Commission européenne avec le chancelier allemand, il a pas participé vendredi dernier un Conseil européen à Prague qui a été largement consacré à la question de l'énergie. La Commission doit faire des propositions, elles doivent nous permettre d'apporter des réponses à hauteur des enjeux lors du Conseil européen des 20 et 21 octobre. Nous avançons dans plusieurs directions. Nous allons mener un dialogue renforcé avec les partenaires qu'ils nous fournissent du gaz. Nous devons faire bloc, alors que la Russie tente de déstabiliser notre modèle démocratique. Nous sommes d'accord pour mettre en place des achats groupés qui nous permettent d'éviter la concurrence entre États membres et compagnies gazières, la Commission va présenter des règles qui permettront aux États et aux entreprises d'agir de concert dans le dialogue avec nos fournisseurs. Enfin, nous avançons vers l'idée d'un plafonnement temporaire du prix du gaz. 2 dispositifs sont à l'étude. Le 1er est un prix plafond pour tout le gaz consommé. Le second est un élargissement à toute l'Europe du dispositif qui a permis de diviser par 3 les prix de l'électricité en Espagne. Ce dispositif ibérique permet de plafonner le prix du gaz servant à produire de l'électricité, ils pourraient utilement servir de base à une mesure européenne. Nous travaillons en parallèle au niveau français, à d'autres mécanismes pour ramener les prix à des niveaux raisonnables. Plus largement, enfin cette crise nous invite à réformer rapidement et en profondeur le marché européen de l'électricité. Nous devons trouver des solutions durables pour offrir aux Européens des prix raisonnables et proche des coûts de production. Ne soyons pas naïfs, les années à venir seront difficiles, notamment en matière d'approvisionnement en gaz. Toutes ces mesures sont donc essentielles pour permettre à notre pays et à l'Europe d'affronter dans la durée, la situation sur le front de l'énergie. Mesdames et messieurs les sénateurs, si nous répondons avec force à l'urgence, nous devons dès maintenant préparer notre avenir. Les énergies fossiles ont des des effets dont nous connaissons les ravages sur la planète, elle nous expose à des fluctuations de prix majeur. Elles sont une source de fragilité dans notre quête de souveraineté nationale et européenne, mais comme nous en sommes dépendants donne dans notre quotidien, nous continuons à les consommer. Nous devons sortir, nous voulons être la première grande nation industrielle à s'émanciper des énergies fossiles. C'est le cap fixé par le président de la République, début février, à Belfort, avant même le début de la guerre. C'est une question de souveraineté car nous serons moins dépendants de l'approvisionnement d'autres pays, nous serons également davantage mettre des prix, c'est un impératif climatique : sortir des énergies fossiles, c'est le levier majeur pour atteindre la neutralité carbone en 2050. C'est une protection pour les ménages, les collectivités et les entreprises à qui nous pourrons offrir des énergies propres et compétitive. Pour atteindre cet objectif, il faut un plan des moyens et des points de rendez-vous. de la Moby ou pardon car c'est de la responsabilité collective que vient le succès. C'est le sens de la planification écologique dont j'ai la charge et c'est ainsi que nous construirons notre transition énergétique. Pour réussir notre stratégie repose sur 3 piliers. La sobriété d'abord une production d'électricité décarbonnée ensuite autour du nucléaire et du renouvelable et enfin le développement de nouveaux vecteurs énergétiques comme l'hydrogène décarboné. Le premier axe de notre stratégie, c'est la sobriété énergétique. Avec les crises que nous traversons et l'appel du président de la République en juillet dernier la sobriété a fait son apparition sur le devant du débat public. La sobriété, ça n'est pas le choix de la décroissance, c'est baisser un peu la température décaler ses usages et éviter les consommations inutiles. Ce sont aussi des actions structurelles comme la décarbonation de notre industrie, comme la rénovation énergétique massif de nos bâtiments ou encore le renouvellement de notre éclairage public. Je pourrais égrener longtemps la liste des exemples, hein, la sobriété c'est efficace et c'est une source d'économie pour tous, État, collectivités, entreprises, particuliers, chacun doit prendre sa part et agir à la hauteur de ses moyens. Sous l'égide de la ministre de la transition énergétique des travaux ont été menés, secteur par secteur pour identifier les économies d'énergie possible sans impacter l'économie. Grâce à ce travail et à la mobilisation de tous, nous avons été en mesure de présenter la semaine dernière un plan de sobriété complet et ambitieux, un plan qui permettra de réduire notre consommation énergétique de 10 pour 100 d'ici 2 ans. J'entends certains se plaindre de l'absence de mesures coercitives, ce plan, c'est la preuve que la responsabilité collective marche c'est notre meilleur chemin pour réussir, j'y crois pour notre transition énergétique et notre transition écologique. C'est de cette manière que chacun pourra identifier les actions les plus efficaces. C'est de cette manière que nos actions pourront remporter l'adhésion. Mais je le répète, la sobriété ne s'arrêtera pas à la fin de l'hiver. Nous visons une baisse de notre consommation d'énergie de 40 % d'ici 2050. La sobriété est une manière de penser et d'agir, qui doit s'inscrire dans la durée, ce plan est donc un point de départ, c'est le 1er pas d'un long chemin. Le 2ème, axe de notre stratégie, c'est le développement du nucléaire et du renouvelable. Le rapport demandé par le président de la République à RTE et remis l'année dernière nous a éclairé sur les différents scénarios possibles. Pour remplacer les énergies fossiles, même si nous consommeront moins d'énergie au global, nous devons produire plus d'électricité pour satisfaire nos nouveaux usages, notamment la mobilité électrique ou les chauffages plus performant, concrètement, nous devons être en mesure en 2050, de produire jusqu'à 60 % d'électricité de plus qu'aujourd'hui. Face à ce défi beaucoup portent des solutions toutes faites. Certains ne jurent que par le nucléaire, d'autres au contraire voudrait fermer nos centrales et ne s'appuyer que sur les énergies renouvelables. Ce sont, au demeurant, parfois les mêmes qui s'opposent à la réalisation concrète des projets. Nous nous choisissons de suivre les experts pas les idéologues nous cherchons ce qui est efficace pour notre production d'énergie bon pour notre économie et protecteur pour la planète, la crise actuelle nous montre l'urgence de la diversification, elle prouve que nous ne devons pas être dépendant d'une seule ressource, elle révèle que dans les moments de tension, même les apports énergétiques que l'on peut juger faible sont parfois décisif, un mixe diversifié est une chance, une protection. C'est pour cela que nous devons avancer sur deux jambes renouvelables et nucléaire. Alors oui nous allons développer massivement les énergies renouvelables. C'est un choix pragmatique car c'est la seule manière de répondre à nos besoins immédiats quand il faut 15 ans pour construire un réacteur nucléaire. Vous avez parlé. C'est un choix écologique car décarbonnées. C'est un choix économiquement rationnel, car la production d'électricité renouvelable permet désormais de dégager des recettes pour l'État. Alors que les moyens de production renouvelable coûté 6 milliards de subventions en 2021 ils rapporteront 10 milliards d'euros en 2022 qui seront intégralement redistribués aux consommateurs d'électricité. C'est un choix de souveraineté aussi parce que nous allons continuer à investir dans des filières industrielles. Nos parcs éoliens en mer en mer, comme celui de Saint-Nazaire ont permis de construire en France une véritable filière. Il en est de même pour le solaire, je souhaite que nous puissions réinvestir pour installer en France et en Europe, la production et l'assemblage des panneaux et développer une nouvelle génération de panneaux solaires. Nous nous sommes donc fixé un objectif : doubler les capacités de production d'électricité renouvelable d'ici à 2030. Nous avons donc d'Aix, décidé d'accélérer le rythme. D'ici la fin du mois vous examinerait un projet de loi qui permet d'accélérer le développement de ces énergies renouvelables, notre objectif est de lever les obstacles administratifs et d'aller 2 fois plus vite qu'aujourd'hui. Notre démarche devra naturellement s'inscrire dans le respect des riverains et de l'environnement. Nous miseront principalement sur le photovoltaïque et l'éolien en mer mais pour réussir, nous aurons aussi besoin de l'éolien terrestre. Je connais votre attention à ce sujet, mais je connais aussi votre sens des responsabilités et je le dis devant vous, nous devons améliorer l'intégration dans les paysages et mieux planifier les installations pour rééquilibrer le développement de l'éolien, sur le territoire et éviter l'implantation anarchique des parcs. Enfin, nous allons aussi promouvoir l'hydroélectricité, nous vous proposerons un nouveau cadre législatif qui permettra de relancer rapidement les investissements dans nos pas dans nos barrages sans passer par une remise en concurrence. En parallèle, nous allons moderniser notre parc nucléaire. Notre 1er défi c'est le devenir des réacteurs existants. Le. Nous prolongerons tous les réacteurs qui réponde à nos standards de sûreté. C'est pourquoi EDF conduit actuellement les études nécessaires avec l'Autorité de sûreté nucléaire pour identifier les réacteurs qui ne pourrait pas être prolongée au-delà de 50 ans. C'est pourquoi, conformément aux engagements du président, nous avons lancé un ambitieux programme de nouveaux réacteurs nucléaires. Le 1er volet de ce programme, c'est la construction de 6 EPR de dont le 1er doit être mis en service à l'horizon 2035. Nous devons faciliter et accélérer le développement de ces projets, notamment en allégeant certaines procédures administratives, c'est le sens du projet de loi sur le nucléaire, qui sera présenté en conseil des ministres début novembre. Je connais aussi la qualité et l'implication des salariés de la filière nucléaire je sais pouvoir compter sur eux, c'est l'engagement et l'arrêt de la responsabilité de chacun que viendra notre réussite. La seconde étape de notre programme nucléaire consiste à étudier la construction de 8 réacteurs supplémentaires. Nous devons notamment donner de la visibilité au secteur pour embaucher et former nos chercheurs, ingénieurs et techniciens de demain. Enfin, le 3ème volet de notre programme nucléaire, c'est l'innovation pour bâtir des réacteurs de nouvelle génération. La prend, la France a pris des engagements forts ainsi avec France 2030, nous avons décidé d'investir un milliard d'euros dans le nucléaire du futur, notamment pour la construction d'un prototype de SMR en moins de 10 ans. Le développement du nucléaire doit s'appuyer sur un pilotage rigoureux et un suivi précis, c'est pourquoi nous avons choisi de reprendre le contrôle à 100 % d'EDF. C'est pourquoi nous allons installer une délégation interministérielle pour le programme de nouveau nucléaire cette délégation sera conduite par l'ancien délégué général pour la l'armement Joël Barre. Son expertise en matière de direction de grands programmes sera précieuse pour garantir notre performance industrielle et le respect des délais. C'est pourquoi, enfin, nous travaillons à nous doter d'une filière nuitées nucléaire plus intégrée et que nous soutenons l'acquisition par EDF des activités nucléaires de General Electric. Mesdames et messieurs les sénateurs, le 3ème, axe de notre stratégie, c'est l'investissement dans les vecteurs énergétiques d'avenir, notamment l'hydrogène au service de la décarbonation de l'industrie des transports et du bâtiment. L'hydrogène Ali transition énergétique et industriel, il permettra une décarbonation massive et efficace de notre économie, même dans les secteurs les plus consommateurs comme la sidérurgie et les mobilités lourde. Il fera émerger une nouvelle filière, avec 100 à 100 50 1000 emplois durables à la clé, il sera un atout précieux pour notre souveraineté énergétique. C'est pourquoi nous voulons faire de la France, le leader de l'hydrogène décarboné nous nous en donnons les moyens via France relance et France 2030, nous allons investir 9 milliards d'euros dans les prochaines années, nous construirons une filière d'hydrogène complète sur l'ensemble de la chaîne de valeur, il y a 15 jours, dans l'Oise, j'ai annoncé un investissement de 2 milliards d'euros, qui permettront de bâtir les dix premières giga factories française. J'insiste sur l'hydrogène mais elle n'est pas la seule filière sur laquelle nous travaillons la décarbonation de notre industrie de nos services et de nos usages passera également par la biomasse par la géothermie par le biogaz et les biocarburants. Nous le savons, certaines industries ne pourront pas toutes électrifiées et devront continuer à utiliser du gaz. Pour elle, le biogaz sera du un levier précieux pour décarboner. Mais le biogaz bénéficiera à notre économie et à nos territoires bien au-delà de l'industrie. C'est une chance pour nos agriculteurs qui pourront y trouver une source de revenus complémentaires tout en valorisant leurs déchets et en produisant des engrais naturel c'est enfin une opportunité pour le développement économique de nos territoires ruraux en créant des autres, des employes locaux et non délocalisables. C'est pourquoi nous nous sommes fixé des objectifs ambitieux pour la méthanisation, nous les soutiendrons, par des mesures législatives et réglementaires afin d'en faciliter et d'en accélérer le déploiement. Enfin, je voudrais dire un mot de l'agrivoltaïsme, dont je sais l'intérêt qu'il porte le Sénat. il n'existe pas aujourd'hui de véritable cadre au développement du photovoltaïque isme sur le foncier agricole et forestier. C'est un problème car cela crée parfois une qu'crut concurrence entre agriculture et production d'énergie, on relève aussi des abus qui nuisent à l'ensemble des filières, cela suscite l'inquiétude dans les territoires, pour autant, cela peut être une source de revenus supplémentaires et un moyen de faire baisser les dépenses des agriculteurs. Je sais qu'une proposition de loi sur l'agrivoltaïsme est en cours de discussion dans cette chambre, je souhaite que nous puissions travailler ensemble pour converger vers une définition commune, notre objectif est d'établir un cadre adapté pour le développement de la filière sur foncier agricole et forestier. Mesdames et messieurs les sénateurs, pour être réussi enfin notre transition énergétique doit être Pont pensée et construite en européen. Nous économies sont interdépendantes nos réseaux sont connectés les uns aux autres, les nations européennes sont nos alliés et nous partageons avec elle des défis et des valeurs. Notre souveraineté énergétique doit donc être européenne. à Versailles, lors de la présidence française du Conseil européen, nous avons franchi un grand pas dans cette direction. Les 27 se sont mis d'accord pour sortir au plus vite de notre dépendance aux hydrocarbures russes et pour accélérer notre sortie des énergies fossiles. C'est une étape historique, la sortie du charbon et du gaz se fera avec l'Europe, c'est ainsi que nous ferons baisser plus massivement notre empreinte carbone, c'est ainsi que nous pourrons donner plus de moyens aux énergies décarbonnées de demain c'est de cette manière que nous pourrons résister au choc énergétique. Mesdames et messieurs les sénateurs, je viens de vous présenter les grands traits de notre stratégie énergétique, c'est le cap fixé par le président de la République depuis le discours de Belfort un cap vers la neutralité carbone et vers la souveraineté un cap qui s'appuie sur la mobilisation et la responsabilité de tous un cake, un cap sur lequel nous allons débattre dans quelques instants. Un débat qui sera suivi de l'action et des faits avec les l'examen dans les prochaines semaines d'un projet de loi sur le renouvelable et d'un projet de loi sur le nucléaire. Après les concertations qui s'engage, sous l'égide de la Commission nationale du débat public, nous pourrons vous présenter la loi de programmation énergie-climat Cadre de notre programmation pluriannuelle de l'énergie. Et pour atteindre nos objectifs, nous devrons avancer avec méthode, en planifiant nos actions en les inscrivant au plus près des territoires et en les pensant en européen. Je veux le dire enfin cette transition énergétique sera radicale et rapide, elles imposent des changements dans nos manières de penser, de consommer et de produire. Je veux conclure en partageant de conviction avec vous. Thierry. D'abord la transition énergétique sera le synonyme d'un meilleur niveau de vie. La sobriété et l'électrification changeront nos usages et nos quotidiens, c'est vrai, mais c'est pour le mieux, elle nous protégerons des chocs énergétiques et des crises à venir, elles permettront de faire baisser les factures en consommant moins nous dépenserons moins je veillerai à ce que la transition énergétique soit une transition juste. Enfin la transition énergétique sera créatrice de croissance et d'emploi, elle sera un levier pour réorienter nos formations et nos compétences vers des secteurs d'avenir, la décarbonation et les rénovations créeront des emplois durables dans de nombreux secteurs, et la transition énergétique appuiera notre réindustrialisation avec de nouvelles filières françaises et européennes, par exemple pour le stockage de l'énergie. La transition énergétique est une nécessité et une opportunité, nous devons pleinement la saisir pleinement la mener, nous y sommes résolus en français et en européen, je vous remercie. Dans la suite de notre débat, je vais donner la parole aux orateurs des groupes premier orateur le président Bruno Retailleau. Pour le groupe Les Républicains. Monsieur Monsieur le Président Madame la première ministre messieurs les les ministres un débat sur la politique énergétique, mais un débat sans vote, à une heure tardive et est-ce bien madame la première ministre à la hauteur des enjeux est-ce bien à la hauteur des gens je compte, on voit bien que, depuis l'été. Tout a été fait à l'envers, on nous a demandé de délibéré au mois de juillet, d'abord sur le principe de la construction d'un terminal méthanier qui va importer si je comprends bien du gaz de schiste américain on a délibéré aussi au mois de juillet sur la réouverture d'une centrale à charbon à Saint-Avold et puis dans quelques jours, on aura l'examen d'un texte sur les énergies renouvelables et puis à la fin de l'année, peut-être en début d'année prochaine sur le nucléaire et puis enfin la stratégie globale on terminera par la politique, une programmation pluriannuelle de l'énergie qui pose le cadre général tout aura été fait, donc à l'envers et dans cette affaire, le Parlement aura eu à délibérer à examiner des textes et une stratégie à la découpe sans voir d'ailleurs cette stratégie en avançant dans le brouillard, alors si j'ose l'expression un débat pour éclairer les Français, peut être, peut être, mais c'est déjà trop tard pour l'hiver parce que les décisions qui n'ont pas été prises qui ont été mal prise il y a quelques années vont produire peut-être je n'espère pas des coupures de courant qui était prévisible, j'ai écrit il y a pratiquement 2 ans un livre dont le titre c'était aurons-nous encore de la lumière en hiver, ce que je veux dire par là c'est que si cet hiver dans quelques mois, nous avions des coupures de courant, c'est pas la faute au Covid, c'est pas la photo de sa rouge c'est pas la faute à je ne sais quoi c'est aussi vos propres décisions, celle du président de la République celle Madame la première ministre aussi qu'on voit vous imputer et il peut pas y avoir de stratégie de politique énergétique sans établir un constat, il peut pas y avoir des remèdes sans partir d'un diagnostic, le constat c'est un constat d'échec et très franchement, je le dis sereinement, calmement, ici, c'est plus qu'un constat d'échec, c'est finalement une sorte de Waterloo énergétique, c'est un Waterloo énergétique parce que il faudra nous expliquer comment un grand pays comme la France, grand producteur grand exportateur d'énergie et notamment d'électricité se retrouve dans une situation où on en vient à manquer de l'électricité si cet hiver et si dès maintenant les Français payent cher leur énergie l'électricité mal il est certes l'argent public malgré certes le bouclier que vous avez rappelé il y a quelques instants, c'est tout simplement parce que l'énergie l'électricité elle est rare et si il est rare, c'est parce qu'on a accompli un bond en arrière d'une trentaine d'années, le niveau de notre production actuelle, c'est le niveau de la production de 1990 alors qu'on est des millions et des millions de Français en plus alors que, on va vers une économie avec des nouveaux usages qui feront appel de plus en plus à l'électricité, c'est ça et vous avez parlé d'EDF voilà un fleuron national qui est totalement fragilisé qui atteindra bientôt sans doute le 60000 et 60 milliards d'endettement fragilisé par un mécanisme, ça n'est pas qu'à vous qu'on le doit d'ailleurs de la reine ou finalement ce fleuron français de l'électricité aura subventionner des concurrents qui, pour la plupart, ne produisent pas un électron hein, bien sûr, bien sûr, mais EDF c'est aussi vous l'avez rappelé un projet d'étatisation, plutôt que de nationalisation, il eut bien mieux valu, à mon avis, ajouter de l'argent frais, c'est-à-dire recapitaliser plutôt que de nationaliser vous nationaliser pour désintéresser les minoritaires mais si vous aviez ajouté cet argent qui va servir à nationaliser pas pour acheter les 16 % de minoritaires mais pour ajouter à la force économique à la puissance financière d'EDF serait vraiment conforté je pense EDF Flamanville, une blessure, mes chers collègues à la fierté nationale, ça n'est pas votre faute Madame la première ministre je sais pas ce que je veux dire, mais c'est une blessure à la fierté nationale à notre ambition, hein, une centrale qu'on devait ouvrir à l'époque, en 2012 qui qu'on a toujours pas ouvert qui devait coûter quelques milliards quand coûtera sans doute plus de deux 3 fois plus pratiquement plus de 4 fois plus, où on doit apporter, faire venir des ouvriers américains pour pour la soudure, c'est une blessure la fierté française, je le crois et je pense que vous le partagez mais ce que j'ajoute, c'est que, en plus de cette blessure aujourd'hui s'ajoute une injustice pour les Français, parce que les Français vont devoir à l'avenir, payer les conséquences des inconséquences de la politique d'Evan Macron les choses sont claires et ça n'est pas la politique de la doudoune qui va vous permettre de vous dédouaner de cette responsabilité, ça n'est pas possible, ça n'est pas monsieur le président d'EDF, à qui l'on doit la décision de fermer en 2017 14 réacteurs nucléaires, ça n'est pas à lui, c'est au président de la République, ça n'est pas non plus au président d'EDF, qu'on doit d'avoir signé un décret d'avril 2020, vous le connaissez, vous l'avez signé avec le Premier Ministre de l'époque, ça n'est pas le président d'EDF, il faut mettre les responsabilités des uns et des autres en face des Verts, des vraies décisions. Et devant cet cet échec en réalité énergétique, il faut revenir en en réalité à ce qui a pu en être les ressorts est-ce que ces décisions ont ont été des décisions fondées sur une vraie stratégie, je ne le crois pas ces décisions, le plus souvent, ont été fondés sur la politique, la petite politique politicienne, Emmanuel Macron et vos gouvernements ont été en quelque sorte les exécuteurs testamentaires d'un qui a eu lieu à l'époque entre Madame Duflot et Madame Aubry pour permettre l'accession au pouvoir de Monsieur Hollande, ensuite il y a eu aussi, bien entendu, la politique de monsieur Macron, avec cette volonté d'avoir monsieur Hulot l'éphémère ministre de l'écologie au gouvernement qui l'a fait, qui lui a fait continuer sur finalement cette cette lancée, c'est la petite politique politicienne, ça n'est pas des décisions qui nous sont tombés de l'extérieur, mes chers collègues, et vous avez beaucoup parlé d'Europe, j'ai été scandalisé lorsqu'ml Macron vous l'avez tous entendu il y a quelques semaines, a voulu justifier la fermeture de Fessenheim, il a justifié. Vous m'entendez bien, la fermeture de Fessenheim en disant, Fessenheim et tu en bordure d'Allemagne, tout près de l'Allemagne à la frontière, or l'Allemagne avait choisi une autre politique et donc évidemment pour fermer les réacteurs et les centrales nucléaires et, par conséquent, il fallait que la France, l'affaire vous pourrez vous faire repasser le ta Verbatim c'est exactement la justification qu'a donné le président de la République et qui est inacceptable, inacceptable et quand je vous entendais parler de l'Europe, je suis désolée, quand on n'a pas de stratégie. La seule stratégie qu'on ait c'est celle des autres, celle de Bruxelles et, derrière, il y avait celle de l'Allemagne, vous en appeler à la solidarité, vous croyez vraiment que l'Allemagne aujourd'hui comme hier, a fait montre de solidarité sur le plan énergétique non mais vraiment, vous pensez vraiment à ce que vous avez dit. Et je ne parle même pas des 200 milliards du boucler énergétique qu'est-ce qui s'est passé, mais moi je suis européen, mais justement, jamais, jamais l'Allemagne n'a cessé, défend ses intérêts, jamais la le, la France n'a défendu vraiment ses intérêts, voilà le problème, voilà le problème, mes chers amis, l'Allemagne s'est mis dans la main de la Russie en achetant peu cher le gaz russe en voulant exporter notamment ses voitures en en et elle a handicapé l'ensemble de l'Europe et nous, on a suivi parce qu'on croit, la solidarité parce qu'on croit au coup fente franco-allemand, moi j'aimerais y croire mais j'attends, j'attends un certain nombre de garanties de nos amis allemands, bien sûr, et aussi de l'Europe, ce qu'on demande un président de la République, il n'est pas président de la République fédérale d'Allemagne, c'est d'abord à Bruxelles de défendre bien entendu les intérêts de la France et des Français, c'est absolument capital alors maintenant, il faut une stratégie, il faut donc une politique énergétique d'abord, je dirais que cette politique énergétique, elle doit. être une constance, une cohérence, elle ne peut pas s'accorder avec le en même temps qui est tout sauf une boussole, sauf un cap pour avoir une politique, une stratégie il faut cette cohérence, il faut cette constance, c'est la première chose, ensuite il va falloir jouer sur l'ensemble des leviers le levier de la production d'abord. Produire de l'offre, le levier de la demande, c'est-à-dire et j'y reviendrai, notamment la sobriété mais pas que et puis aussi la tarification les prix. J'ai commencé par les prix puisque je critiquais la politique européenne, vous vous souvenez très bien, on était dans la même position, ou à ma place et vous à la vôtre, c'était au mois de juillet, vous veniez de prononcer un discours de politique générale je vous répondais et à l'époque je vous avez indiqué, mais Madame la première ministre, pourquoi ne faites-vous pas ce que l'Espagne et le Portugal viennent de faire. Et c'est ce que vous nous proposez aujourd'hui mais on a pratiquement perdu plus de 3 mois, la tarification européenne est une tarification stupide, sans doute, qu'elle a avantagé l'Allemagne elle dessert la France, le président de la République, je l'ai écouté tout à l'heure s'il y avait de débat mais qu'une, chers collègues, il y avait un débat ici à neuf heures et demie, puis un autre débat à la télévision avec le président République qui débattait de la stratégie énergétique de de la France, qu'est ce qui nous a expliqué le président de la République, il a dit, bien sûr, il faut décorrélés le prix de l'électricité, du gaz, mais fallait le faire maintenant, il y avait même des dispositifs qui nous permettaient de le faire deux reprend la main, nous Français, mais à partir du moment où on n'essaie toujours de jouer une forme de solidarité européenne, mais qui n'est pas de la solidarité parce que la solidarité c'est une réciprocité, on est dans la naïveté, on est dans la netteté, donc je vous demande, nous vous demandons de sortir bien entendu de découpler une fois pour toutes, le prix de l'électricité du prix du gaz, il faudra sans doute aller plus loin, moi je vous demande et avec mon groupe que vous puissiez mettre fin à la suspension des accords en tout cas du cadre et des tarifs réglementés qui doivent s'achever au 30 juin prochain je pense qu'il faut en sortir si vous voulez un vrai bouclier, ça n'est pas seulement de l'argent public qu'on doit sur les ménages ou sur l'économie, il y a des décisions à prendre, il faudra repousser j'ai pas entendu un seul élément de langage sur ses tarifs réglementés, c'est fondamental, de même que il faudra autoriser EDF et les pousser une fois le pic tarifaires à conclure des contrats de long terme, l'Europe s'est souvent posée au nom de la concurrence pure et parfaite, mais au nom de cette concurrence pure et parfaite que de problèmes n'avons-nous pas connu depuis les années 2000 2010 démantèlement d'EDF tarification du gaz, donc moi je veux bien la solidarité européenne, mais à la condition que cette solidarité ne mène pas dans le mur, mes collègues,

le télétravail, bien sûr, ce sont des leviers et ça c'est pas une politique. ça n'est pas une politique, expliquez-moi comment en 20 ans en 20 ans nous avons autant régressé en matière de flexibilité de la demande de la sobriété, il y a 20 ans, l'effacement notamment au auprès des particuliers, je vous parle pas des entreprises, ça nous rapportait jusqu'à 6 gigawatts 20 ans après 06 en 20 ans on a divisé par 10 on a divisé par 10 parce que honnêtement Tempo et j'en suis un usager ça marche pas bien ce que j'ai vous proposées ou est-ce que vous en êtes, il faut un grand dispositif national d'effacement rémunéré et volontaire de l'énergie ou est-ce qu'on en est, il faut accorder là encore la volonté et la raison et les nouvelles technologies soyons modernes Madame la première ministre et puis je terminerai sur la la production sur l'offre, il faut produire plus une une énergie qui est quatre critères qui soient abondante qui soit décarbonnée qui soit pilotable et qu'qui soit bon marché parce qu'on ne réindustrialiser pas la France, mes chers collègues, si il y a pas cette énergie bon marché compétitive cet élément qu'on a malheureusement abandonné, il faut donc bien entendu, revoir la PPE déplafonner déplafonner, vous l'avez pas dit l'énergie dans le mix de l'énergie, notamment nucléaire 2ème chose prolongée tant que la sécurité, le permet, les réacteurs nucléaires, il faudra assurer de la visibilité à EDF, je veux que vous engagez ce soir pour que EDF on préserve son unité, pas de projet ou de projets démantèlement sur 10 ans, dites-le nous ce soir, franchement Madame. La première ministre des tôles nous

l'Allemagne a montré mes chers collègues, que quand on investit jusqu'à 40 % l'énergie en terme de renouvelable, il faut aussi investir dans du fossile, c'est ce qu'a fait l'Allemagne, hé bien non, nous on veut aussi une énergie décarbonée oui sur le pilotable oui, bien sûr, sur l'énergie renouvelable, mais il faut aussi, là aussi, savoir raison garder et enfin je crois que mes chers collègues, il faudra là encore une volonté, je terminerai mais la ma Premier Ministre et je conclurai monsieur le Président, en indiquant qu'il y a quelques quelques années en 2017 celui qui vous a nommé avait eu un slogan, un de ses slogans c'était penser printemps, il semble qu'après une crise sanitaire et une crise géopolitique et même Macron découvrent que l'hiver, ça existe aussi que être souverain être souverain ça pèse aussi ce que nous vivons aujourd'hui, c'est ce que le progressisme a oublié mes chers amis, c'est la souveraineté nationale qu'est l'horizon indépassable des nations, c'est cela et ce que je souhaite, c'est que vous cette souveraineté énergétique pour le pouvoir d'achat des Français et pour la réindustrialisation de notre pays, merci madame le. Journaliste merci merci merci Monsieur le Président. Je vais donner la parole à notre collègue Franck Montaugé dans le groupe socialiste, écologiste, les républicains. Monsieur le Président Madame la première ministre, messieurs les Ministres, chers collègues, la politique énergétique nationale nécessite cohérence, constance et résolution, le moins que l'on puisse dire, c'est que depuis trop longtemps, les gouvernements n'ont pas eu cette exigence pour notre pays, je passe sur les tergiversations et les atermoiements du président de la République en matière de politique nucléaire alors qu'il nous faut rapidement actualisées la ASN baisser la PPE, vous nous présentez. Ces jours ci, un projet de loi technique au demeurant nécessaire centré sur les procédures, quel est votre logique, pourquoi ce saucissonnage, alors que les Français et leurs élus ont besoin de lisibilité, de partage des objectifs pour s'engager eux aussi dans la transition énergétique, nous devons collectivement réussir une transition de civilisation parce que c'est de ça qu'il s'agit avec la fin de l'usage des énergies fossiles carbonés et les mises en Oeuvres de modèle de développement fondé sur la notion de durabilité dans un cadre de justice sociale et d'équité, mais cet impératif de long court beaucoup trop négligée jusqu'ici, malgré de nombreuses alertes doit être conjugué avec des réponses immédiates et financièrement accessibles aux besoins actuels des entreprises et de tous nos concitoyens, les Français doivent être soutenus, davantage qu'ils ne le sont par les mesures que vous proposez et ils ne comprennent pas que la France ne puisse pas les aider, comme l'Allemagne s'apprête à le faire pour son peuple, avec un plan de 200 milliards d'euros sur les marchés de l'énergie, des mesures structurelles fortes doivent être aussi prise mais j'y reviendrai, enfin nos propos au regard des enjeux climatiques et environnementaux des techniques de production énergétique disponible de leurs impacts identifier et de leur coût des incertitudes et risques qu'elle présentent le débat de ce soir doit prendre appui sur les données scientifiques et les études techniques dont nous disposons, c'est donc dans le cadre du dernier rapport du GIEC et de l'étude de RTE sur les futurs énergétiques de la France a eu raison de 1050 que je présenterai les analyses et les préconisations de mon groupe, le rôle majeur que doit, selon nous, et dans l'intérêt général, jouer le groupe EDF sera réaffirmé et nous vous questionne sur le projet qui est le vôtre pour ses trente entreprises d'ici peu 100 % public au nom de mon groupe, je souhaite que vous nous disiez ce soir, quelles sont les hypothèses et les orientations que vous retenez pour engager sans tarder le pays vers le futur énergétique dont il a besoin pour lui-même et à l'égard de ses partenaires européens et mondiaux, dans la perspective de neutralité carbone à horizon 2050, la future loi énergie-climat devra confirmer la trajectoire d'extinction des sources d'énergies décarbonnées cela signifie scène du pétrole enfin des gaz d'origine fossile et substitution de l'électricité et du gaz décarbonés à ses ressources dans la SNPC l'électricité représenterait 55 % de l'énergie finale consommée, contre 25 % aujourd'hui, cet objectif est-il le vôtre ou antennes des vous le réviser et si c'est si c'est le cas à quel niveau, dans cette hypothèse, à 55 % d'électricité dans les jeunes énergie finale consommée RTE propose de 6 scénarios du plus sobre à 555 TWh hein au plus élevé à 754 TWh lié à une production en quantité d'hydrogène à décarboner et à la réindustrialisation profonde de notre économie, l'électrification plus ou moins rapide des filières hein et des usages existants constitue également un critère déterminant de la production électrique nécessaire à partir de ces scénarios quel mix de production énergétique décarboné entendez-vous proposer au Parlement pour la prochaine mise à jour de la PPE en cours, les scénarios de RTE recouvre en fait des choix de politique industrielle, très différent du 50 % de nucléaire au 100 % renouvelable. Madame la première ministre, vous l'avez dit, le président de la République a décidé il y a peu, après avoir donné il y a quelques années, des orientations inverse de commander 6 réacteurs EPR2 et de lancer les études pour 8 EPR de et EDF a engagé le programme grand carénage de prolongation des réacteurs nucléaires existants sous le contrôle de l'ASN, à partir de ces décisions, faut-il comprendre que le gouvernement s'engage résolument dans le sens de mix électrique à 50 % d'énergies renouvelables 50 % de nucléaire, pour la clarté de notre débat et la compréhension de vos propositions, quels sont les facteurs qui ont conduit à ce choix pour mon groupe le mix énergétique doit résulter d'une approche pragmatique s'inscrivant bien entendu dans l'objectif du 0 carbone en 2050 incertitudes et risques au pluriel, doivent être pris en compte dans les choix à opérer par exemple au regard des difficultés rencontrées sur de nombreux territoires pour développer des projets éoliens photovoltaïque ou de méthanisation l'accélération du nombres de projets nécessaires au scénario à très forte proportion d'énergies renouvelables, nous paraît de plus en plus problématique, j'ai dit que que dans le scénario à 100 pour 100 d'énergies renouvelables, il faut multiplier par 21 la puissance installée en photovoltaïque et par 4, celle de l'éolienne terrestre hein de fauteuils photovoltaïque supplémentaires, il faudrait aller 10 fois plus vite ses rythmes sont très supérieurs à ce qu'ont fait nos partenaires européens les plus actifs depuis plus de 10 ans en sommes-nous capables, je vous pose la question, autre incertitude dans le domaine du nucléaire l'affaiblissement en France et de cette filière industrielle au cours des décennies passées, je ne parle pas ici de l'exploitation, mais de la construction, les difficultés techniques rencontrées aujourd'hui ont conduit à des interrogations quant à la capacité de mener à bien les programmes de prolongation de la durée de vie des réacteurs existants ou de construction et de mise en service dans les temps impartis de nouveaux réacteurs annoncé l'analyse doit aussi intégrer les coûts complets de réalisation, c'est-à-dire les coûts de production d'acheminement et de flexibilité nécessaire au fonctionnement du réseau en toutes circonstances l'impact environnemental des installations de production, notamment en ce qui concerne les sols dans un contexte de. Que la loi énergie-climat a laissé ni fait ni à faire et il nous faut aussi prendre en compte les émissions de gaz à effet de serre, un cycle de vie des systèmes électro-électrique envisageable dans une perspective hautement souhaitable de souveraineté énergétique renforcer les risques liés aux approvisionnements, ainsi que l'existence de filières industrielles nationales doivent être intégrés, vous l'avez évoqué la question de l'emploi local, pour la construction, mais aussi plus encore pour l'exploitation doit traite prise en compte et orienté le choix du mix, s'il fallait faire le choix d'un scénario RTE, les critères d'évaluation que je viens d'évoquer nous amènerait à faire le choix d'un mix, à 50 50 50 nucléaire à 50 renouvelable nous considérons cependant que la situation énergétique dans laquelle se trouve notre pays des Panama des conséquences de la guerre, Anne, Ukraine, je tiens à le souligner, justifie que le gouvernement pousse tous les curseurs dans le sens d'un développement accéléré de tous les modes de production d'énergies décarbonnées pour réussir la transition énergétique hein, situation d'incertitude, voire de risques comme je viens de le dire, hein, il faut que nous nous donnions des marges en matière de puissance installée, nous devons industrialiser les procédures de réalisation des projets de la concertation publique à la mise en oeuvre, c'est fondamental de l'État aux collectivités locales en passant par les comités régionaux de l'énergie Les S trois heures ENR dans l'adaptation aux besoins doit être revu, comment allez-vous mettre en ligne les acteurs sur quels principes repos concret repose votre planification à à ce stade, le projet de loi d'accélération l'énergie renouvelable nécessaire ne ne pourrait pas à la hauteur des enjeux et les difficultés rencontrées sur les territoires, dans ce cadre et pour que l'agriculture contribue à la production énergétique renouvelable française sans réduire sa fonction nourricière première une définition de l'agrivoltaïsme devra être légiférer comme le Sénat s'apprête d'ailleurs à le faire, nous attendons de connaître la position du gouvernement également sur ce point, nous devons aussi aborder avec vous, la question du devenir du groupe EDF du projet que le président de la République et le gouvernement Antoine de lui donner dans ce contexte énergétique pour le moins instable et cela ne date pas de la crise ukrainienne dans les faits et le départ du PDG Lévy attestent après avoir passé 5 ans à ne prendre aucune décision à la hauteur des enjeux, le président de la République et ces gouvernements sont restés muets sur le rôle qu'ils entendent faire jouer à EDF, dans le contexte extrêmement que nous lui connaissons aujourd'hui, jamais depuis sa création en 1946 cette grande entreprise nationale n'a été autant affaibli par défaut de pilotage politique pertinent, c'est à se demander si tout cela n'est pas voulu significativement l'ancienne présidente de la creux disait lui-même il est je crois dans votre gouvernement aujourd'hui depuis 10 ans, EDF a été la vache à lait de l'État, fin de citation je rajoute que les personnels dévoués aux missions d'intérêt général de l'entreprise n'y sommes pour rien, la responsabilité et politique et exclusivement politique, nous souhaitons que vous vous en expliquiez dans le cadre de ce débat, madame la ministre Madame la première ministre pardon, pouvez-vous nous présenter les conséquences institutionnelles et juridiques de l'OPA que vous avez lancé le statut actuel de l'entreprise est-il amené à évoluer vers un épique par exemple quel rôle exact l'État actionnaire unique pardon va-t-il jouer une OPA ne fait pas un projet industriel, quel est votre projet industriel, social et environnemental pour EDF, avez-vous et ses grandes demain souhaitables renoncer au découpage de l'entreprise, comment financer, vous les investissements d'EDF nécessaires au grand carénage aux énergies renouvelables, ainsi qu'aux réseaux de distribution et de transport et les faits et les flexibilités qui vont avec : pouvez-vous nous expliquer comment et dans quel cadre juridique, vous allez financer le nouveau nucléaire commandé par le chef de l'État, ce financement sera-t-il réalisé dans le cadre du groupe EDF ou Andorre et si oui comment, quelle place, entendez-vous donner à la production hydraulique, comment envisagez-vous de préserver dans la durée, le caractère public de ce parc de production je voudrais aborder la dimension européenne du sujet, si le est une prérogative nationale des États membres, le marché de l'énergie et placé sous la responsabilité de l'Union européenne, il y a là une contradiction interne qui explique en grande partie les difficultés que subissent de nombreux consommateurs français et européens et ça et ça ne date pas de la crise ukrainienne, quelles propositions le gouvernement français va-t-il porter au niveau de la Commission européenne et de la puissante DG concurrence pour que le marché et les prix payés par les consommateurs particuliers et industriels reflète au plus près les coûts complets sur long terme des mix énergétiques nationaux, nous souhaitons que les tarifs régulés de l'électricité perdure et que ceux du gaz soit maintenue également au-delà de la date de suppression annoncée, nous vous demandons de faire en sorte que les petits consommateurs obtiennent des prix stables dans le temps et que les chefs d'entreprise et la et de la visibilité en matière de prix de l'énergie sur le moyen et le long terme, je vous remercie. Je vais donner la parole à notre collègue Denis Saint-pour le groupe de l'Union centriste. Vous avez la parole. il nous faut établir ce que nous sommes en droit d'attendre d'un système énergétique, premièrement, de la sécurité et j'entends derrière ce concept sécurité d'approvisionnement afin d'éviter délestage rationnement et black-out, la 2ème exigence, c'est le maintien de notre souveraineté, notre système énergétique doit dépendre le moins possible de puissances étrangères, surtout quand ces dernières sont potentiellement instable ou hostiles, troisièmement pour atténuer le changement climatique en cours, notre système énergétique doit tendre vers la neutralité carbone à l'heure actuelle, force est de constater qu'il présente malheureusement des lacunes sur les 3 tableaux la plus visible en ce moment, concerne l'insécurité d'approvisionnement avec le spectre d'une pénurie d'énergie qui ressurgit pour l'électricité, cela tient notamment au vieillissement des centrales nucléaires quant au gaz, il fait désormais défaut aux Européens, du fait de la guerre en Ukraine, même si la France en souffre moins que nombre de ses voisins, ces déficiences nous rendent par conséquent dépendant de l'étranger, qu'il s'agisse de notre voisin allemand pour l'électricité en période de pointe ou bien de la Norvège et du Qatar pour le gaz, enfin notre mix énergétique n'est pas assez décarboner car plus de 60 % de nos besoins énergétiques sont encore satisfaits par du gaz et du pétrole en cela il est vrai que nous faisons mieux que bien d'autres pays mais c'est encore largement incompatibles avec les objectifs fixés par l'accord de Paris sur le climat, il nous faut donc réformer notre système énergétique à la fois pour répondre aux enjeux immédiats et pour garantir les générations futures, à court terme, le gouvernement semble avoir bien saisi les enjeux depuis plusieurs mois, il était effectivement nécessaire de sécuriser l'approvisionnement en gaz de notre pays en trouvant de nouveaux fournisseurs, ce qui a permis de remplir nos stocks au maximum avant l'hiver à moyen terme, il faudrait toutefois envisager de produire ce gaz sur le sol national, par exemple, laver la méthanisation, de même il fallait organiser la sobriété pour réduire les tensions sur notre système électrique, c'est l'intérêt du plan dévoilé jeudi dernier, rappelant qu'en la matière, les efforts doivent concerner autant l'État et les entreprises que les particuliers et les collectivités territoriales, enfin je salue Madame la Ministre votre mobilisation constante et celle de votre gouvernement auprès de la Commission européenne pour qu'elle propose des solutions collectives aux États membres, c'est à ce niveau que les actions seront le plus efficaces en matière énergétique, car c'est à l'Union européenne de régler le problème central posé par cette crise, celui de la formation du prix de l'électricité, ce dernier correspond au coût marginal du dernier opérateur connecté au réseau, or aujourd'hui ce dernier opérateur, ce sont les centrales à gaz dans le coût de production tire l'ensemble des prix vers le haut, aussi faut-il découpler au plus vite le prix de l'électricité de celui du gaz, pour ce faire de voix existent, soit par le haut, soit par le bas, par le haut, c'est-à-dire en créant un grand service européen de l'énergie publiques et monopolistique hélas cela relève actuellement de l'utopie, nous n'arrivons déjà pas à nous mettre d'accord sur la taxonomie. L'autre voie la plus réaliste est une sortie par le bas, c'est-à-dire une forme de rats renationalisation du système, c'est ce qu'on fait l'Espagne et le Portugal, avec l'aval de la Commission européenne, ils ont ainsi le droit durant un an de déconnecter le prix du gaz, de celui de l'électricité, de fait, cela leur réussit tandis que fin août, le prix du mégawattheure était de 660 euros en France et en Allemagne, il n'était que de 240 euros en Espagne et au Portugal, cette dérogation leur a été accordé pour 2 raisons : ils sont très peu interconnecté avec le reste de l'Europe, et ils ont une électricité très décarbonés symétriquement, cela signifie que l'on doit envisager la solution ibérique pour les pays européens dans l'électricité est déjà largement décarbonés comme la France, la situation actuelle ne peut en effet plus durer une fois nos centrales, remise en ordre de marche notre situation énergétique serait meilleur en faisant cavalier seul avait le monopole d'EDF plutôt que dans le marché de l'électricité communautaire dans le même ordre d'idée, l'ouverture du marché de l'énergie n'a pas donné des résultats satisfaisants revenir dessus nous permettrait de supprimer cette absurdité qu'est la reine, ce dernier a été une belle aubaine pour des opérateurs qui se sont comportés comme de simples négociant engrangeant des profits sur l'argent du contribuable investi dans les centrales, il est temps désormais d'arrêter de considérer l'énergie comme une simple marchandise et la prendre pour ce qu'elle est réellement un bien public de première nécessité, à ce titre, il convient de s'interroger sur la pertinence d'un éventuel retour aux tarifs réglementés de vente de l'électricité et même du gars à plus long terme, c'est d'une vision stratégique dont nous avons besoin, telle que celle présentée par le président de la République dans son discours de Belfort en février dernier, cette stratégie repose sur le triptyque sobriété nucléaire et renouvelables, nous ne pouvons qu'y souscrire mais lorsque l'on regarde de plus en détail ce beau tableau, les choses se compliquent singulièrement premièrement les projections relatives à la sobriété nous semble irréaliste, certes nous pouvons renforcer nos efforts sur de nombreux plans tels que l'isolation des bâtiments où l'consommation mais 40 % de besoins énergétiques en moins en 2000 Tarente alors que nous saurons un peu plus nombreux et 20 % plus riches si la croissance moyenne n'est que de 1 pour 100 d'ici à cette date, qui peut y croire, c'est pourtant sur une telle anticipation que repose la stratégie nationale bas-carbone et tous les scénarios de RTE, en adoptant des hypothèses plus réalistes, ce sera déjà une très belle performance d'arriver simplement à maintenir et non augmenter nos besoins énergétiques d'ici à 2040, mais dans ce cas de figure, ce n'est pas 60 % d'électricité en plus qu'il nous faudra produire au tournant du siècle, mais le double ou le triple, c'est bien pourquoi les annonces faites jusqu'ici en matière de nucléaire, même si elles vont incontestablement dans le bon sens nous semblent bien trop insuffisantes à Belfort, le président de la République a déclaré qu'aucun réacteur un état de produire ne doit être fermé, mais le plan de fermeture de 12 réacteurs d'ici à 2035 et toujours en vigueur, va, va-t-il enfin être officiellement abandonné dans l'affirmative, va-t-on prolonger nos réacteurs au maximum, c'est une question clé car le nombre d'EPR à construire en dépend de plus aucun plan de développement de SMR n'a été annoncée alors que le petit nucléaire semble une solution d'avenir prometteuse, enfin, la recherche et l'innovation dans le nouveau nucléaire semble relancé, mais à quelle fin précisément fermeture du cycle du combustible, réacteurs de 4ème génération thorium il faut un plan et des objectifs, enfin pour ce qui est des renouvelables, je ne veux pas ici empiéter sur les débats qui seront les nôtres lors de l'examen du projet de loi ENR, mais je peux déjà dire que le groupe de l'Union centriste, plaidera en faveur de l'essor de l'agrivoltaïsme de la géothermie et de la biomasse, plus globalement, chacune des 3 volets du plan français, va se heurter un grave problème de ressources humaines il faut pas former dès maintenant de vrais professionnels du nucléaire, des réseaux électriques intelligents de l'isolation des bâtiments et des ENR, avons-nous un plan de formation digne de ce nom pour faire face à ses besoins, si oui, il nous faudra le connaître les événements autant que le sens de l'histoire nous invite à un Big bang énergétique montrons-nous à la hauteur de ce rendez-vous, je vous remercie. Merci, cher collègue. La parole est maintenant notre collègue Didier Rambaud pour le groupe Rassemblement des démocrates progressistes et indépendants. Merci, Monsieur le Président Madame la première ministre, messieurs les ministres, mes chers collègues, l'énergie, occupe une place dans le débat public, qu'elle n'a sans doute jamais eu auparavant et pour cause : guerre en Ukraine contexte d'inflation tensions autour des carburants dérèglement climatique autant de de défi qui nous rappelle que l'énergie abondante et à bas prix n'existe plus, préparer l'avenir, tout en apportant des réponses à l'urgence, c'est au fond Madame la première ministre la double stratégie de la France pour répondre à ces défis majeurs d'une part, à court terme pour sauver notre approvisionnement, d'autre part à long terme pour assurer la souveraineté énergétique de la France et sa neutralité carbone pour ce qui est de notre approvisionnement, cela n'a échappé à personne, dans un contexte d'inflation Poutine utilise l'énergie pour faire la guerre, nous faisons face, comme nos voisins européens à une situation extrêmement délicate, le gouvernement fait donc le choix d'impulser une nouvelle solidarité européenne agir collectivement pour s'entraider et s'alimenter en électricité pour l'hiver, agir avec solidarité pour que nous évitions les coupures en matière de gaz, il a été décidé d'alimenter nos stocks auprès d'autres fournisseurs, nous permettant ainsi de les remplir à hauteur de 99 par ailleurs, le Parlement a voté en juillet dernier, l'accélération du projet de terminal flottant au large du Havre des décisions prises avec rapidité à la hauteur de la crise géopolitique et qui nous permettront de passer le prochain hiver nous l'espérons, avec le moins de difficultés possible néanmoins, soyons lucides : si l'approvisionnement de nos stocks et nécessaire : réaliser des économies d'énergie n'en reste pas moins indispensable et cela de manière collective, à commencer par l'État qui doit être exemplaire, sans oublier les collectivités, les entreprises et l'ensemble des Français, c'est tout l'esprit du plan de sobriété que vous avez présenté jeudi dernier Madame la première ministre un plan qui prône l'incitation et la responsabilité collective, pas de privations, ni de textes de loi tout simplement des gestes de bon sens, des gestes du quotidien que parfois nos aïeux faisait déjà sobriété ne signifie pas décroissance et tant que nous le pouvons, saisissons l'option de la sobriété choisie plutôt que d'attendre la sobriété subit, reconnaissant au passage qu'il s'agit aussi d'une opportunité pour lutter contre le gaspillage énergétique et la surconsommation, le groupe RDPI soutient totalement cette stratégie cette stratégie qui ne doit pas nous faire perdre de vue que face à l'urgence, l'État doit aider les acteurs les plus en difficulté, je rappelle que le gouvernement comme le Parlement n'ont pas été inactifs en la matière, pensons au bouclier tarifaire sur les prix de l'énergie qui sera reconduit en 2023 pensons également aux 430 millions votés d'euros votés dans la loi de finances rectificative en juillet dernier à destination des collectivités qui permettront à une part significative du bloc le communal d'avoir un peu d'air après le quoi qu'il en coûte, qui a permis de sauver notre économie désormais face à l'inflation, les Français, les PME et les collectivités resteront protégés, c'est la promesse de ce gouvernement, toujours à l'offensive pour conserver nos emplois et notre pouvoir d'achat mais, chers collègues, notre pays n'en reste pas moins confronté à 2 défis de taille : assurer la souveraineté énergétique et atteindre la neutralité carbone d'ici 2050, rien ne serait pire que de penser une fois l'hiver passé, que la crise énergétique deviendrait un mauvais souvenir à oublier les défis liés à l'énergie seront au coeur des débats politiques des années à venir renforcer notre souveraineté, c'est d'abord investir dans le mixte énergétique prendre conscience que l'éolien en mer, le photovoltaïque, l'agrivoltaïsme et l'hydraulique sont autant d'énergie renouvelable qu'il nous faut développer en concertation avec les élus locaux, renforcer notre souveraineté c'est aussi admettre que le nucléaire doit prendre toute sa part dans le mixte énergétique aujourd'hui le nucléaire représente environ 70 % de la production électrique française avec un modèle basé sur l'électro-nucléaire, il serait déraisonnable de s'en passer, les Allemands ont souhaité faire ce choix, et ils sont aujourd'hui largement dépendant du gaz, bien entendu, la part du nucléaire doit être complémentaire avec celle des énergies renouvelables, mais le nucléaire est une force historique, nous devons la conforter, toujours est-il que notre parc est vieillissant et et requiert beaucoup de maintenance, on ne peut pas se satisfaire que 26 réacteurs sur 56 sont actuellement indisponible, nous récoltons aujourd'hui les fruits de mauvais arbitrage passer la nationalisation d'EDF est un mal nécessaire pour réarmer et consolider notre ancien fleuron un projet de loi sera justement présenté dans les prochains mois pour simplifier les procédures et permettre de faciliter la création des nouvelles générations d'EPR renforcer notre souveraineté c'est aussi réduire les délais administratifs pour accélérer sur les énergies renouvelables, un projet de loi permettra en novembre 2 débattre en profondeur de ces questions, mais regardons les choses avec lucidité le tout nucléaire ne fonctionnera pas et le tout ENR ne fonctionnent aura pas davantage pour atteindre nos objectifs, nous devons diversifier, réduire les délais administratifs, simplifier les procédures libérer du foncier encourager le partage territorial de la valeur, autant d'objectifs qui seront au coeur du projet de loi d'accélération des énergies renouvelables, encore une fois mon groupe sera au rendez-vous de ce travail parlementaire, renforcer notre souveraineté exige également de se réindustrialiser, c'est l'objectif du plan France 2030 avec 2 milliards d'euros, dédié à l'innovation dans les énergies renouvelables et le nucléaire, la France peut se donner les moyens de construire par exemple le premier avion bas carbone, mais la France peut également être en mesure de réindustrialiser avec des énergies décarbonnées énergie tels que l'hydrogène ou encore le gaz provenant de déchets organiques mon département l'Isère est un territoire à ce sujet, qui illustrent bien la production de ce type de gaz 9 sites hein jette injecte déjà du biométhane dans les réseaux, dont 2 sont en chantier et devrait en injecter d'ici la fin de l'année, enfin notre souveraineté requiert une solidarité européenne ne confondons pas souveraineté et protectionnisme en matière d'énergie, nous devons penser en Européens l'histoire nous rappelle que l'ancêtre de l'Union européenne était la Communauté européenne du charbon et de l'acier, créée par 6 États en 1951 dont la France, il ne fait aucun doute que les mécanismes européens de tarification doivent être réformés, nous devrons décorrélés le prix de l'électricité, l'électricité, du prix du gaz, les défis sont techniques et complexe, mais nous savons que le gouvernement met toute son énergie pour convaincre nos voisins européens, Nietzsche pensais que l'Europe ne se fera qu'au bord du tombeau, le moment est peut-être venu de créer une nouvelle union européenne énergétique, mes chers collègues, les spécialistes, les ingénieurs, les scientifiques nous rappelle aussi une réalité de bon sens, l'énergie la plus propre et celle que l'on ne consomme pas alors je ne prône pas le le retour à la bougie, ben, je suis convaincu qu'en matière d'énergie, comme dans le milieu du sport notre boussole doit être le collectif encouragé le collectif pour pour la mobilité encourager le collectif en matière de choix énergétiques encourager le collectif enfin en matière de sobriété, se dire que si tout le monde s'y met avec esprit de responsabilité et de solidarité, l'État, les collectivités et les entreprises, et nous tous, en tant que citoyens, nous nous donnerons les moyens d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Merci, cher collègue. La parole est à notre collègue Fabien. Pour le groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste. Monsieur le Président Madame la première ministre, messieurs les ministres, mes chers collègues, nous vivons une période critique décisive charnière, l'urgence est là pour notre économie pour les entreprises, les collectivités, les citoyennes et les citoyens, la crise énergétique que nous vivons est un défi, et elle va s'inscrire dans la durée la situation nous oblige avec lucidité dans une optique constructive, nous devons étudier comparer et débattre des moyens de notre politique et souveraineté énergétique surtout, nous devons nous montrer capables d'une vision d'ensemble nous ne résoudrons pas cette crise énergétique en l'abordant segments par segments, comme vous nous le proposez un texte cet été sur les dérogations réajustements puis un sur les renouvelables qui va venir, un autre sur le nucléaire, un autre qu'on apprend sur l'hydroélectricité dès ce soir, et enfin une loi de programmation pluriannuelle de l'énergie, on ne sait quand et au passage la re-étatisation d'EDF par amendement au contraire nous avons besoin d'une vision d'ensemble, au risque de subir et de revivre des crises car ce que nous traversons aujourd'hui cette envolée des prix ces menaces de Blackout, ce n'est pas qu'un simple et malheureux empilement des conjonctures c'est l'obsolescence d'un système énergétique tout entier qui est en train de s'écrouler, il y a une dimension conjoncturelle, c'est indéniable, le déclenchement de la guerre en Ukraine, bien sûr, puis était digne d'un cataclysme climatique lui aussi lourd de conséquences sur la production électrique, les besoins climatisation décuplé en Espagne, et avec eux la comme sommation énergétique du pays, des sécheresses record, comme vous l'avez dit, partout en Europe et des rideaux inédite pour les barrages français qui produisent 12 % de l'énergie du pays, nous avons connu un niveau d'eau historiquement bas, le tout dans un contexte de mise à l'arrêt de la moitié du parc nucléaire, dont une partie n'était pas prévu une somme de facteurs qui se conjuguent et qui échappe à notre emprise directe et immédiate, mais ce que nous maîtrisons et ce qui nous appartient, c'est la décision politique et ce que nous voulons, ce n'est pas un État actionnaire qui gère comme le privé mais à État volontariste et stratège qu'a une vision d'avenir, parce que l'emballement des prix de l'énergie que nous connaissons aujourd'hui, c'est un résultat Direct du marché européen de l'énergie et de plus de 20 ans de libéralisation du secteur lié le prix du gars, c'est l'électricité, nous conduit à cette situation. Ou le prix payé par des États et par les consommateurs ne reflète en rien le mix électrique national quand le kW/h atteint 1000 euros, comme il l'a fait cet été, nous ne parlons pas d'une réalité matérielle, mais d'un résultat spécule Athis et artificiel, les Français, les Européens ne paient ni le coût ni le prix de l'énergie, mais celui de l'Europe libérale et des traders, il suffit de regarder le fonctionnement, celui d'un prix de l'énergie qu'on meurt à tous les États membres les usagers paient le même prix que leur pays investi dans le nucléaire dans les renouvelables ou qu'il soit resté dépendant des énergies fossiles, faisant le bilan de ce mécanisme en France, seuls 7 vers 7 % de la production électrique dépendent du gosse, rien ne justifie que les cours de l'électricité, dopé par les prix du gaz se répercute sur nous avec une telle force allô chercher une sortie temporaire du marché européen, emboîtant le pas de nos voisins espagnols et portugais qui ont fait valoir que non, ils n'ont pas à subir les cours du gaz qui ne reflète aucunement leur mix énergétique, d'ailleurs, je suis très heureux que vous disiez ce soir que vous en êtes d'accord, il faudra juste le dire à votre secrétaire d'État chargé de l'Europe qui hier en audition devant la commission européenne du Sénat, a dit le contraire, nous avons en France 92 % de notre mix électrique issue du nucléaire de l'hydraulique du photovoltaïque du solaire et de l'éolien 92 nous avons réduit nos importations de gaz et notre dépendance aux énergies fossiles, nous sommes donc légitime à porter cette demande sur la scène européenne, alors Madame. La première ministre, je ne vous apprendrai rien en vous disant que nous avons des débats politiques mais je tiens à vous le dire, si vous décidez d'engager cette bataille. Nous l'amèneront à nouveau à vos côtés, entendons-nous bien, je ne parle pas d'interrompre toute carte interconnexion. Car il faut garder de la solidarité européenne, il s'agit là de réformer le système européen en profondeur ou dans le sortir, mais c'est un chantier qui prendra des années, nous pouvons donc obtenir une dérogation dans les prochaines semaines, si nous nous battons, car nous n'avons pas des années pour agir, les dégâts sont déjà là d'abord pour nos collectivités territoriales, les factures explosent 30 % en moyenne, pour certaines, nous en sommes à 150 % dans mon département de millions d'euros pour Noisy-le-Sec, idem pour Neuilly sur Marne et près de 30 millions pour le département des arbitrages intenable sommes déjà en préparation, quelles que soient nos couleurs politiques, augmenter les impôts locaux renoncer à des investissements majeurs comme la rénovation thermique des bâtiments ou fermer des services publics, nous devons créer un bouclier tarifaire réel immédiat ah rétablissant les tarifs réglementés de l'électricité pour toutes les collectivités territoriales et baisser la TVA à 5 5 pour tous les usagers, quant à la fin des tarifs réglementés de vente du gaz en juillet 2023, c'est un grand danger dans la période il faut empêcher coûte que coûte cette extinction, c'est une nécessité absolue, qui concerne aussi les entreprises électro-intensives avec l'inflation des prix de l'énergie, nous savons pertinemment que l'emploi sera la variable d'ajustement des fermetures sont déjà envisagées ou du chômage partiel, comme chez Duralex et Arc International Madame la première ministre, je pose la question quel sera le coût du chômage partiel pour l'État : sommes-nous vraiment dans un scénario préférable au rétablissement des tarifs réglementés pour tout le monde, y compris les artisans et commerçants, comme les boulangers, c'est que l'été Hervé sont préférables au bilan social qui est à craindre, nous allons traverser au moins 2 ans de crise et les prix, nous redescendrons jamais ah enfin nous avons 12 millions de personnes qui sont en situation de précarité énergétique combien de plus vont basculer combien d'impayés vont tomber, il y a une urgence sociale pour les 2 prochaines années il faut interdire les coupures de tous les fournisseurs, et pas que d'EDF et garantir une puissance minimale à 3 kilowatts contre, hein, aujourd'hui, il faut des actions fortes dans l'immédiat, couplée à une planification c'est un impératif qui pose la question d'EDF Madame Lamy la première ministre je salue l'organisation de ce débat, pardonnez-moi. Merci, mais je regrette que le Parlement ne soit pas associé sur une question aussi essentielle que la rue étatisation d'EDF, le débat est légitime une raie étatisation oui mais pour quoi faire, si c'est pour faire un. Projet recule de qui viendra séparer les activités et à m'ouvrir aux capitaux privés, pour nous, c'est non et sans attendre 2025. Il faut sortir de la reine, ce système qui n'a fait qu'enrichir les opérateurs alternatifs et des PC EDF car si nous défendons un grand service public de l'énergie avec monopole public c'est précisément. Que la crise actuelle nous en offre une démonstration, le secteur privé et inapte sur cette question, d'autres crises nous le prouverons dans les années à venir, nous devrons investir 10 milliards d'euros pour la sortie des énergies fossiles, il nous faut d'ailleurs impérativement nous extraire de la charte européenne de l'énergie, ce traité de pleins pouvoirs, multinationale qui leur permettra de réclamer des milliards à des États pour défendre leur investissement dans les énergies fossiles et maintenant caduque, nous défendons enfin le développement d'un mix électrique, avec des investissements dans le nucléaire de nouvelle génération et dans les énergies renouvelables, que pour notre part nous n'opposons pas. Nous avons besoin d'une programmation de l'énergie réelle, concrète, qui reposent sur des indicateurs fiables et avec une entreprise publique solide qui a les capacités d'investir et pour cela nous devons sortir l'énergie du secteur marchand et en faire un bien commun de toute l'humanité, je vous remercie. La parole est à notre collègue Franck Menonville pour le groupe, les indépendants républiques et territoires. Vous avez la parole. entre le printemps 2020 et le 1er septembre 2022, les prix de marché ont été multipliés par 3, pour le pétrole, 5 pour le gaz et 40 pour l'électricité, comment on s'nous sommes arrivés là, la reprise économique après le vol le plus fort de la pandémie, a généré des tensions sur les marchés, avec le retour de l'inflation, le 24 février en envahissant l'Ukraine, Vladimir Poutine a déclenché un conflit entraînant, entre autres, une flambée sans précédent des cours de l'énergie en en se servant ainsi du gaz comme moyen de pression, l'Europe qui était dans un état de dépendance vis-à-vis des hydrocarbures russes est aujourd'hui dans une situation difficile, ce qui nous annonce un un hiver particulièrement compliqué, il faut le dire, la France est structurellement moins dépendante du gaz russe que l'Allemagne et, notamment, qui a renoncé au nucléaire, la situation de la France semblait meilleur en théorie,

Cette année nous serons pour la première fois, importateur d'électricité parce que nous avons pas su anticiper et préserver notre parc pour illustrer cela, le 21 juillet 2022, 2022, RTE a apporté en moyenne plus de 7000 mégawatts sur le marché spot européen, soit 15 % de la consommation nationale, une certaine idée de l'écologie pou poussait donc pour la réduction, voire la disparition du nucléaire aujourd'hui notre filière va mal et mal en point et fragilisé, nous devons tout faire pour conserver nos savoir-faire et garantir son avenir à Saint-Nazaire le 22 septembre dernier le président Macron a esquissé alors que nous sommes au pied du mur, l'accélération de la stratégie nucléaire de la France, Encore, nous étions les champions du monde de l'énergie nucléaire civile, nous disposions d'une autonomie et nous exportations même notre excédent électrique, nous avons baissé la garde en menant des politiques contradictoires, guidé par des choix idéologiques mon sont manquons souvent de réalisme, je pourrais citer Ségolène Royal, qui souhaitait baisser de 75 à 50 % la part du nucléaire à horizon 2025 une orfèvre en matière de géopolitique et de planification énergétique ne devrions-nous pas Madame la première ministre réviser cet objectif qui Uzice encore dans la loi, à horizon 2035 nous sommes bientôt en deux en 2023 alors même que nous le savons, les besoins d'électricité seront croissant à la longue liste qui nous conduit à la situation actuelle, on peut ajouter l'abandon du jeu du du projet de centrale Superphénix de traitement des déchets nucléaires en 1997, le projet Astride portant pourtant lancée en 2010, abandonné en 2019 100, programme de recherche alternatif, fermant ainsi la porte à de nouvelles avancées technologiques, la décision de fermeture de Fessenheim prise sur le sous la présidence de François en nous obligeant aujourd'hui dans notre région Grand-Est à réouvrir une centrale à charbon, je ne parle paraît pas de l'affaiblissement continu des capacités financières d'EDF

il me semble que les précédents grand ministère de l'écologie et du Développement durable n'avait pas naturellement dans leur ADN, la capacité de planification énergétique et industriel, nous attendons beaucoup de la constitution de ce nouveau ministère de la transition énergétique qui semble aller dans le bon sens, notre pays a besoin d'un grand ministère de l'énergie et de l'industrie, par ailleurs, force est de constater qu'on a affaibli dans notre pays le le le dans notre pays donc le pilier du nucléaire sans pour autant atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés dans la PPE en matière de développement d'énergies renouvelables en effet la les complexités administratives rendent le déploiement des ENR difficile et beaucoup trop long sur par rapport à nos voisins européens, notre bouquet énergétique a besoin tant du nucléaire que des énergies renouvelables, les projets de loi qui sont, qui que vous avez annoncé aujourd'hui doivent absolument pouvoir devoir y répondre, il faut travailler sur tous ces leviers, il n'est pas acceptable d'attendre plus de 10 ans pour voir naître un projet éolien ou solaire porté et voulu par les territoires sur nos territoires, pratiquement le double des pays européens qui nous entourent la crise à laquelle nous devons faire face rend cependant criant le besoin d'un changement structurel de notre politique énergétique française, notre économie est déjà touché par la crise économique, il faut bien surveiller à ne pas fragiliser davantage notre issue économique dans le cadre d'un éventuel délestage il faudra absolument être en mesure de de protéger et de prison prioriser la capacité productive actuellement, force est de constater qu'en France, de plus en plus d'usines tourne au ralenti à cause des prix de l'énergie, nous nous sommes sommes sur nos territoires tous alerter sur la situation complexe voire intenable dans le temps en matière d'industrie d'artisanat et quelquefois d'accès d'agriculture également beaucoup de nos chaînes de valeur sont mises en péril par des importations plus compétitive la crise énergétique est en train de porter un coup dur à notre industrie au moment où ou mon mouvement donc nécessaire de réindustrialisation dans la France a besoin nos collectivités territoriales, nos industries, nos entreprises ainsi que les ménages français, déjà fortement affecté subissent d'ores et déjà les conséquences économiques de cette crise énergétique, les inquiétudes qui nous remonte du terrain sans grandissante, la France a mis beaucoup de peu à mis bien en place, donc un bouclier tarifaire afin d'aider, donc les ménages à faire face à l'envolée des prix de l'énergie, ces mesures nécessaires ont un coût et sont à un coût important et pourtant elle demeure incomplète au regard des disparités des situations rencontrées sur le terrain, l'Europe doit au plus vite, trouver des solutions, il faut penser différemment la politique énergétique européenne et plus précisément le marché intérieur européen d'une énergie, nous devons donc découpler le prix de l'électricité de celui du gaz, vous l'avez annoncé pour conclure : nous devons bâtir une véritable stratégie de long terme,

et la promotion d'économie d'énergie, reposant sur la recherche, le développement de technologies économes sur la rénovation énergétique deuxièmement le défaut, autant que possible des énergies renouvelables et troisièmement la relance du nucléaire autant que nécessaire, en accentuant nos savoir-faire technologique, mes chers collègues, il n'y a pas de place pour l'idéologie et le dogmatisme, nous devons porter une vision de long terme, répondant besoin croissant de notre demande d'électricité décarbonnée et ainsi vers l'aller vers la sortie programmée des dernières. Merci mon cher collègue. Donner la parole maintenant à notre collègue Jean-Pierre. Pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen. Monsieur le Président Madame la première ministre, messieurs les ministres, mes chers collègues, le gouvernement a présenté la semaine dernière son plan de sobriété, on peut se féliciter de cet encouragement, même tardif à la sobriété, il aura encore fallu une situation de crise et une urgence tant économique que sociale pour que l'État pressent le pas, nous n'aurions sans doute pas pu éviter la crise, mais ses effets auraient été moins explosif, la réduction de la consommation énergétique de 40 % d'ici 2050 pour atteindre la neutralité carbone se fera désormais sur une trajectoire de là dont la pente sera bien raide, nous sommes là pour débattre, pour partager les constats mais aussi réfléchir à des solutions pour éviter que ce désastre situation ne se reproduise Bordeaux, donc la question de manière ascendante et comme l'aurait dit mon collègue Fabien Gay, la situation de nos concitoyens, tout d'abord, malgré les multiples demandes et alerte des acteurs locaux, qu'ils soient publics ou associatifs, et en dépit des annonces successives d'un grand plan national de rénovation énergétique des bâtiments, force est de constater que le compte n'y est pas issu d'un département où les températures ne sont pas toujours clémente et où l'habitat individuel notamment minier comptent parmi les moins bien isolés malgré un gros rattrapage ces dernières années, je peux mesurer au quotidien combien il reste à faire et pour les habitants concernés, c'est la double peine, nous savons que ceux qui sont dans les habitations les plus énergivores sont également ceux qui vivent des situations économiques et sociales parmi les plus dramatiques, il suffit de parcourir les documents de bilan des dossiers des fonds vérité logement pour s'apercevoir du niveau de précarité, de fragilité, de nombreux ménages le chèque énergie constitue certes une aide mais elle ne peut agir que comme un pansement face aux perspectives d'augmentation des tarifs qu'on nous annonce et la baisse progressive du bouclier tarifaire, j'ai déjà interpellé l'État à plusieurs reprises sur la question du reste à charge des aides proposées par l'Anaes, il reste dissuasif pour un trop grand nombre de nos concitoyens, c'est le même problème que pour le coût de l'essence, les personnes modestes ont souvent des véhicules anciens plus consommateurs que de carburant, là encore, j'ai contesté en son temps, quand j'étais le rapporteur sur le bonus-malus, madame la ministre à l'époque du de la suppression du dispositif d'accompagnement financier à l'achat de véhicules hybrides et de sa limitation à l'achat de voitures électriques dont les tarifs, même avec une aide reste prohibitif pour beaucoup regardez l'explosion du prix de la Zoé nous faut là aussi réfléchir désormais à un vaste plan de conversion notre parc automobile et d'accompagnement des ménages les plus modestes à l'acquisition de véhicules plus propres, deuxièmement, la situation de nos collectivités, maintenant j'ai interrogé la semaine dernière, votre ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, sur l'augmentation alarmante des coûts de l'énergie pour nos collectivités et l'inquiétude des élus face à cette situation, insuffisance prévisible de l'enveloppe ouverte en loi de finances rectificative imprécision quant aux modalités de mobilisation de ce fonds inadaptation des critères, repoussant l'obtention des fonds au mieux à l'été 2023 sur toutes ces questions, le ministre a s'est voulu rassurant, il a promis des réponses rapides, espérons-le, mais surtout ces réponses devront être adaptés, ne pas être soumises à des critères trop restrictifs, désormais, seuls 8000 communes au lieu de 20 mille semblent pouvoir prétendre à l'enveloppe de 430 millions d'euros dernièrement une nouvelle explicative adressée en fin de semaine dernière par le secrétariat de monsieur Attal fait état de trois critères cumulatifs à remplir, on complexifie on renforce, au final, ce sont peut-être encore moins de communes qui pourront émarger à ce dispositif, faut-il rappeler ici les déclarations récentes de la ministre en charge des collectivités, évoquant une réévaluation de l'enveloppe jusqu'au milliard si nécessaire une preuve s'il en était besoin, la ville vulnérabilité de nos collectivités à ce rythme, les 430 millions ne sont peut-être même pas consommé, je vous ai entendu dire Madame le 1er Ministre peut-être des avances avant la fin de l'année, je vais utiliser un mot à la mode, chiche, n'oublions pas que les collectivités sont des acteurs majeurs dans le dynamisme de l'économie locale grâce notamment leur investissement la crise énergétique hypothèque nombres de projets reportés ou parfois même abandonnées, y compris ceux orientée sur le développement des énergies renouvelables une transition donc toute faite avec le projet de loi à venir sur l'accélération des énergies renouvelables, un texte qui, sous couvert d'accélération comporte des dispositions qui doivent nous interpeller, difficile d'entente retards imputables à l'État lui-même qu'il se donne même pas les moyens humains et financiers d'instruire le dossier serve de cochon pour remettre en cause les principes de la consultation citoyenne, ainsi que la protection de la biodiversité et des paysages, mais Madame Pannier-Runacher à qui je souhaite un prompt rétablissement, nous a rassuré, il y a une dizaine de jours qu'donc quand même que nos procédures administratives sont parfois inutilement lourde et retarde les projets de ce point de vue, la qualification de raisons impératives d'intérêt public majeur prévu dans le texte constituerait un véritable recul en termes de démocratie participative et un danger pour la préservation de notre environnement, sauf à ne l'utiliser par exemple que sur la rénovation des anciens parcs éoliens en augmentant la puissance et sur le fond, il serait illusoire, voire mensonger de laisser penser que cette accélération des ENR sur la solution à nos difficultés, le recours aux énergies naturelles ne pourra en aucun cas être une solution à la demande d'énergie, mais ce qu'elles sont par nature intermittentes. En outre, il est dommage que le texte fasse l'impasse sur un point important, celui de la constitution de véritables filières du renouvelable acté le principe d'une accélération de synergies renouvelable est une chose mais créer les conditions de sa réussite nécessite de sécuriser toute la chaîne, afin de la pérenniser, d'autant plus que l'éolien est aujourd'hui recyclable à plus de 97 il faut garantir un soutien financier durable et prévisible de l'État, assurer une politique de formation efficiente travail allez l'attractivité de ces filières lutter efficacement contre les malfaçons avec une politique de Label pour autant au sein du RDSE, nous saisirons ce texte par nous sommes parce que nous sommes conscients de l'urgence, mais en tentant d'en corriger les excès et pour y introduire des améliorations, considère le développement de ces énergies renouvelables et la préservation de la nature, les sujets sont techniques complexes en matière d'énergie, je pense à l'hydroélectricité absorbe du projet de loi sur l'accélération des ENR, je pense aussi à l'agrivoltaïsme je pense, enfin la filière du biogaz et au gaz vers elle aussi grande oubliée du projet de loi sur les ENR, ce matin même un un problème existe je posé à Arras, la première Pierre de État Centre de méthanisation des déchets ménagers de la communauté urbaine d'Arras et je ne comprenais pas que les boues de la station de la purgation à côté, ne pouvait pas être métallisé, alors qu'en Allemagne les boues de stations de d'épuration sont méthane Isablle plus, plus de 15 ans toutes les pistes doivent être étudiées et l'ensemble des acteurs écoutez, si on veut atteint les objectifs fixés dans les déclarations du président de la République à Belfort et repris dans le plan sobriété, je reste convaincu que la solution réside dans le dans la diversité du mix énergétique, l'occasion de soulever un autre incohérence, à mon sens, pourquoi mobiliser un projet de loi différents sur le volet nucléaire de notre approvisionnement énergétique, il nous faut travailler dans l'articulation des modes de production, il aurait été plus logique de traiter la question énergétique dans un seul et même texte après avoir discuté de la programmation pluriannuelle énergétique, comme l'a dit le président Retailleau tout à l'heure, projeté un développement du parc nucléaire est une chose, les sommes ici sur du moyen voire du long terme, sur, surtout si l'on se réfère aux douloureux épisode du 1er EPR assurer le redémarrage de la moitié de notre parc aujourd'hui maintenant en est une autre Madame la première ministre, vous nous avez donné des assurances et pour nous réellement compter sur ce renforcement avant l'hiver, la rue nationale sur d'EDF représente aussi une opportunité pour reprendre en main notre avenir industriel et Roulers celui nucléaire mais à quelle échéance et à quel prix s'accompagnera-t-elle d'un retour aux tarifs réglementés pour la collectivité, si la France ainsi que d'autres États ont pris position en faveur d'un découplage entre le prix de l'exercice du gaz, la réforme du marché européen de l'électricité pourra-t-elle être mise en place avant que les conséquences, nos entreprises ne constituera ce désastre. Je vous remercie, merci mon cher collègue, donnait la parole à notre collègue Daniel seulement pour le groupe écologiste solidarité et territoires. On avait la parole. Monsieur le Président Madame la première ministre, mes chers collègues, en septembre 2021 déjà 12 millions de Français ne pouvait pas se chauffer, comme il le souhaitait, un an après, à l'approche de l'hiver, l'Europe traverse une crise économique et géopolitique qui mettent en lumière les lacunes systémiques de nos sociétés en matière d'approvisionnement énergétique, cette crise questionne en profondeur notre modèle de consommation et valide, ne vous en déplaise, le projet que les écologistes depuis des années. Les stratégies à mettre en place pour sortir des énergies fossiles, atteindre la neutralité carbone en 2050 et ainsi respecter les objectifs de l'accord de Paris sont plus que jamais attendu et urgente, elles doivent être à la hauteur des enjeux historiques. L'abondance énergétique a une enfin nous le savons depuis des décennies, notre développement assis sur l'extractivisme se heurte à la finitude de la planète et à la saturation de son atmosphère en polluant aujourd'hui en matière de politique énergétique pour respecter nos engagements climatiques différentes options sont sur la table. Au préalable, je voudrais réaffirmer qu'il n'y a pas de production d'énergie parfaitement propres, excepté celle que l'on ne consomme pas et j'y reviendrai concernant la production, la seule option qui permette une transition soutenable et durable est un mix énergétique que nous appelons de nos voeux et qui n'a pas changé : nous défendons le déploiement massif de nos énergies renouvelables vers le 100 pour 100 en 2050 et en parallèle la sortie programmée du nucléaire nous revers Liens Dron sur le sujet en fin d'année, oui, une France 100 % renouvelable en 2050 est techniquement possible sans mettre en péril la sécurité d'approvisionnement, comme le souligne l'un des scénarios de RTE scénario totalement crédible, comme le rappelle son président, nous devons y aller parce que c'est l'énergie la plus propre, la plus sûre, la plus résilientes et la moins chère, vous l'avez rappelé Madame la première ministre, cette énergie est aujourd'hui extrêmement compétitive et rentable nous Loïc occasion de défendre ce déploiement massif est indispensable dans les futurs véhicules législatif mais en attendant, les retards pris pour engager la France sur les rails de la transition énergétique et l'absence d'anticipation des gouvernements successifs sont particulièrement graves, ils sont la cause de notre dépendance aux énergies fossiles, ainsi que de la crise sociale profonde qui en découlent, que de temps perdu, les énergies renouvelables, ce sont les énergies des territoires, les grands projets comme les plus petits, comme l'illustrent les centaines d'initiatives partout en France, les habitants, les élus locaux souhaitent prendre leurs responsabilités face aux crises, il souhaite aussi créer des circuits courts, de l'énergie et de nouvelles solidarités locales, c'est pourquoi les politiques publiques doivent renforcer la concertation l'implication, l'investissement des habitants et des collectivités locales dans les projets. La dynamique de l'énergie citoyenne rouage essentiel de l'essor des renouvelables à condition de changer de braquet dans les modes de soutien qui lui sont consacrés, donner également davantage de moyens aux collectivités locales dans la mise en oeuvre de la transition écologique est indispensable et doit aller bien au-delà du fonds climat que vous, doté de 2 milliards. Rappelons que les collectivités territoriales compétentes EPCI Région se sont vu transférer de nouvelles compétences sans aucun transfert de moyens par conséquent les plans et schémas en faveur de la transition énergétique ne pourront être mis en oeuvre et risque de rester en grande partie à l'État d'intentions. Au-delà du financement, l'action des collectivités implique également de développer des moyens d'ingénierie dans les territoires et d'accompagner le secteur privé, avançons pour structurer réellement cette mise en mouvement généralisée des territoires en faveur de la transition énergétique, c'est tout le sens du service public des énergies renouvelables que nous défendons depuis longtemps avec le groupe écologiste solidarité territoire service public qui permettrait de planifier les politiques publiques en la matière. Permettez-moi, en fin d'accès mon propos sur un autre sujet majeur de notre indispensable transition la planification de la sobriété, c'est le seul moyen de réguler notre consommation afin de respecter les limites planétaires, tout en réduisant les inégalités qu'on soit clair, la sobriété, ce n'est pas un instant Goran temporaire pour passer l'hiver, c'est le principe d'organisation économique et sociale nécessaire pour respecter l'accord de Paris et sauvegarder pour l'indique dot l'espèce humaine, parce que la sobriété sans égalité c'est l'austérité pour les plus pauvres, nous défendons une sobriété juste. Près de 2 ans après avoir raillé le modèle Amish le gouvernement a finalement dû se résoudre à l'évidence en s'engageant dans un plan de sobriété mais sans réelle contrainte sur le secteur privé, y compris sur les plus gros pollueurs sans mesures pérennes structurante, ce plan n'est clairement pas à la hauteur des enjeux, une série de petites mesures de bon sens, mais au bon vouloir de chacun, comme d'habitude Madame la première ministre vous n'allez nous vous n'avez même pas regardé la première des mesures contraignantes qui figurait dans le programme du président-candidat puis dans votre déclaration de politique générale, rendre obligatoire l'indexation de la rémunération des dirigeants des grandes entreprises sur le respect de leurs objectifs environnementaux nous sommes encore bien loin de la planification écologique promise pendant la campagne présidentielle, j'ajouterai qu'il n'y a pas de solution à la crise énergétique que nous ne connaissions 100 lutte contre les injustices et sans remise en cause des privilèges de certains alors que tant d'entre nous, subissent déjà au quotidien une sobriété contraintes tous les comportements et pratiques de consommation des plus riches ne soit pas réguler cadré est injuste et inefficace. Rappelons qu'aujourd'hui les disparités en matière d'émission de carbone sont colossales quand Monsieur Bernard Arnault prend son jet-privé et émet 160 16 tonnes de dioxyde de carbone en un mois, soit l'équivalent de 17 ans d'empreinte carbone d'un Français moyen oui le déni de justice et la vertigineux, sans recherche d'une répartition juste des efforts à accomplir toute politique ou recommandations de sobriété énergétique sera vécu comme une forme d'austérité contraignante et injuste par les plus pauvres et précaires ce plan manque donc sa cible et alors qu'on compte plus de 5 millions de passoires thermiques impossible à chauffer l'hiver et rafraîchir l'été, ce plan ne prévoit que 100 millions d'euros de plus pour financer ma rénovent, soit à peine 4 % d'augmentation moins que l'inflation des coûts de la des coups de l'isolation et ce, alors que ce dispositif dysfonctionne n'est pas assez doté ni suffisamment efficace, ce rapport fait donc l'impasse sur l'essentiel : stopper les productions superflus, réduire les inégalités, financer les services publics et l'isolation des logements, il ne reprend rien la force subversive et politique de ce concept de sobriété et reste aveugle à la nécessité d'un changement de paradigme concernant nos modes de consommation, pourtant la sobriété est compatible avec le bien-être et même susceptible de la croate, plutôt qu'une perte de confort, la transition vers une sobriété juste assurera les besoins fondamentaux se loger, se nourrir, se déplacer dans une meilleure équité sociale, le respect que nous devons aux générations futures et l'indispensable prise en compte du vivant sur la Terre. En conclusion, la politique énergétique que nous défendons, c'est le droit à l'énergie pas au gaspillage que chacune et chacun ait accès à une énergie abordable, aujourd'hui et demain à une énergie qui ne nuise ni aux écosystèmes, ni à la santé, les mesures à prendre d'urgence pour passer l'hiver sont en réalité les mêmes que celles qui doivent nous permettent de préserver une planète vivable et faire durablement baisser le prix de l'énergie, réduire et partager produire l'indispensable, voilà la philosophie des écologistes discutons planifions repolitiser c'est il doit être avant tout un choix de société Madame la première ministre, vous nous avez vous vous êtes engagé tout de suite à reconstruire une filière photovoltaïque dépêchez-vous car Photowatt détenues par EDF est en train de mourir, il est grand temps de remettre en place des filières dans l'énergie renouvelable en France, vu le fiasco de la filière nucléaire, nous ne pouvons que faire mieux. Merci, Monsieur Stéphane Ravier pour la réunion administrative des sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe, vous avez la parole. Oui, le meilleur pour la fin pour vous réveiller mes chers collègues. Monsieur le Président Madame la première ministre, mes chers collègues Madame la première ministre c'est curieux ou vous êtes exprimée dans cette assemblée, comme si vous étiez encore en mesure de décider de quoi que ce soit, or depuis le traité européiste de Lisbonne à la politique énergétique et des États membres est une compétence partagée avec la Commission européenne, par la suite, notre pays, chef de file historique de la filière nucléaire aurait dû imposer ses vues à ses partenaires, mais les gouvernements successifs ont fait preuve de naïveté et de faiblesse en succombant à l'assaut de 3 force la première, celle de l'Allemagne qui avait fait le choix de la dépendance au gaz russe et qui gagnèrent le bras de fer pour imposer des énergies renouvelables dans les textes et objectif européen celle de l'écologie aussi punitive que médiatique piloté à distance par les grands lobbies américains ça le du dogme de la concurrence libre et non faussée utilisée pour sabrer notre fleuron EDF selon Madame la première ministre vous n'en êtes pas directement responsable mais vous assumez la filiation avec ceux qui nous ont entraînés dans cette folie, ce dont vous êtes responsable, c'est de continuer à nous imposer ses énergies prétendument renouvelables contre la démocratie locale par une circulaire de septembre dernier, vous exigez des préfets qu'casse les PLU dans les cas des communes mentionnerait l'interdiction d'implanter des éoliennes de plus vous préférez limogé le PDG d'EDF, après qu'il ait pointée vos responsabilité dans la situation actuelle, le limogeage devenant une véritable méthode de gouvernement, c'est pourtant EDF qui a racheté au printemps dernier les turbines nucléaires d'Alstom vendus en 2014 à l'américain General Electric par un certain Emmanuel Macron ce n'est pas Jean-Bernard Lévy qui a procédé à la fermeture idéologique et injustifiée dans la centrale nucléaire de Fessenheim c'est vous et vous en étiez fière, en France, on n'a pas de gaz mais on a des idées, la sobriété et le col roulé, vous venez de déclarer vouloir sortir des énergies fossiles, mais vous avez réouvert cet été la centrale à charbon de Saint-Avold, vieille de 71 ans, l'abandon de notre souveraineté énergétique nous a rendu tributaire de l'étranger, c'est pourquoi, en voulant sanctionner Vladimir Poutine votre Europe s'est déshonoré en signant des accords gaziers avec l'Azerbaïdjan finançant ainsi par nos impôts, la guerre menée contre l'Arménie, il faut le dire et le répéter, le nucléaire est notre force économique et écologique, contrairement à l'éolien qui saccagent nos paysages pour une production énergétique dérisoire dérisoire et au solaire qui sont toutes 2 des énergies intermittentes nécessairement couplés aux centrales à gaz et à charbon le grand carénage en cours est un grand plan de modernisation de la filière nucléaire pour le, pour le moment, victime d'un sous-investissement chronique, le nucléaire représente l'avenir, un avenir d'indépendance énergétique, il ne faut pas non plus oublié de protéger notre filière hydroélectrique décarbonés actuellement menacé de libéralisation, il ne manque d'entretien Madame la première ministre ou vous êtes dans le domaine énergétique, qui n'est pas question de croyances mais de pragmatisme et de réalité, je rappelle que la France n'est responsable que de 1 % des émissions de gaz à effet de serre à l'origine du réchauffement climatique, je vous invite donc à vous dépolluer l'esprit des prêches des talibans verdoyant et à tirer les enseignements de vos erreurs, plutôt que d'en faire supporter les conséquences aux Français.

Monsieur le président, Mesdames, messieurs les sénateurs Madame la première ministre merci pour ce débat qui, dans l'ensemble. Ah traité je pense de l'essentiel, c'est-à-dire de l'avenir de l'avenir de nos filières industrielles de l'avenir de notre production énergétique de l'avenir, au fond de la souveraineté française et n'en déplaise à Monsieur Ravier également de la souveraineté européenne, mais j'ai quand même entendu ici ou là quelques critiques sur le bilan quelques critiques sur la politique nucléaire de la France, y compris quelques critiques osé sur le bilan du gouvernement précédent, et de notre président de la République et donc je vois souhaiterait puisque on souhaite ensemble faire le bilan du nucléaire, prendre un peu de recul et revenir à la réalité de ce qui est aujourd'hui l'état des centrales nucléaires en France et de leur histoire, la réalité, ça a été dit un certain nombre de fois sur tous les bancs, c'est que pour faire durer les centrales nucléaires, il faut les entretenir. Et la réalité aussi. C'est que des investissements massifs dans les centrales nucléaires. Qui nous explique sans doute une grande partie de la de la situation d'aujourd'hui, c'est au début des années 2000 qu'elle a, qu'elle avait lieu, on n'a jamais autant désinvesti dans les centrales nucléaires françaises que sous les quinquennats de Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy. Et c'est pas moi qui le dis, c'est la Cour des comptes dans un rapport de 2012 et à l'époque, vous le savez sans doute, puisque vous avez lu le rapport de la Cour des comptes comme moi. La disponibilité des centrales s'est effondré entre 2005 et 2009. Ensuite, vous le savez aussi le choc pour le nucléaire, ça a été l'accident de Fukushima en 2011 qui a conduit l'ensemble des États à revoir leur politique nucléaire: le Japon bien sûr. Le Japon, bien sûr, la Belgique, qui revient sur sa politique de l'époque, l'Allemagne qui n'en est pas revenu et qui a fermé la plupart de ces centrales, je pense qu'il n'reste que trois aujourd'hui, sur les 35 initial et même la France à l'époque, s'est interrogé, je vous rappelle que ni le président Nicolas Sarkozy a décidé d'abandonner le projet d'EPR de Penly, en 2011 et je le comprends suite suite à l'accident ah j'ai compris que certains voulaient tuer le père, moi je fais le bilan de la politique énergétique de la France Monsieur le Sénateur, C'est évident. 11 ans après l'accident de Fukushima. La France avait 58 réacteurs, nous en avons aujourd'hui 56, oui nous en avons fermé de. Mais aujourd'hui, la France est un des seuls grands pays industrialisés qui a gardé le cap sur le nucléaire, et ça, au fond, on doit peut-être à l'ensemble des gouvernements qui ont tenu le choc malgré des sous-investissements malgré, malgré un accident historique et qui fait qu'aujourd'hui on a fait, bah, ce qui nous permet d'investir encore davantage la réalité, la réalité c'est que le ministre de l'Économie, Emmanuel Macron, c'est lui qui a sauvé Framatome, la réalité c'est que le ministre de l'Économie et c'est lui qui a sauvé Areva, la réalité c'est que le ministre de l'Économie et mal un cran, c'est lui qui a recapitalisé EDF qui avait été trop longtemps sous-capitalisées, la réalité c'est que le président de la République, dès qu'il est arrivé, il a revu l'objectif de 50 % de nucléaire pour 2025 pour le repousser de 10 ans à horizon 2035, la réalité c'est que quand nous avons protégé les Français vous allez Français avec le bouclier énergétique, la réalité c'est que nous avons aussi protéger EDF et que nous avons pris sur le Denier public le poids de cette protection, la réalité c'est que c'est le président de la république aujourd'hui, vous l'avez dit à de Belfort en janvier de la de de cette année, qui a annoncé la création là la la

Ce qui m'amène à parler de notre projet pour EDF, puisque maintenant on peut se projeter vers l'avenir, le bilan, j'espère, étant en partie soldé, parler de ce projet de la reprise d'EDF, de la renationalisation d'EDF qui a été annoncé, qui va mettre mise en oeuvre d'ici la fin de l'année, la réalité c'est qu'il ne s'agit en aucun cas d'un démantèlement d'EDF, je pense qu'on n'a jamais évoqué cette possibilité, la réalité c'est qu'il y ait une reprise en main industriel et opérationnel de notre opérateur national la présidente Prima s'en souvient sans doute nous étions ensemble en juin 2018 pour visiter l'EPR de Flamanville, le président Hervé Morin était là également la présidente Barbara Pompili nous étions avec le ministre, Sébastien Lecornu et on nous a expliqué à l'époque que l'EPR de Flamanville commencera à produire ses premiers électrons, janvier 2019 oui, la réalité c'est que père femme en ville, c'est une déception énorme, il a été lancé en 2000, les gouvernements successifs l'allez confirmer certains du bout des lèvres, d'autres avec plus d'ambitions et qu'on n'a pas réussi, je le regrette, a livré la marchandise la réalité aujourd'hui, c'est qu'on a besoin de reprendre en main avec une direction opérationnelle les opérations industrielles et opérationnel de notre grand opérateur national afin qu'ensemble nous puissions à nouveau en être fier, on nationalise EDF pour lever un financement à bas Bakou et pour financer les projets de nouveau nucléaire ont nationaliste pour mettre en place une quasi-régie qui permettra à l'État de garder les barrages, je vois ça, que vous êtes sensible et de réinvestir dans ses barrages, on veut qu'on EDF continue à investir durablement et plus massivement dans les ENR, la réalité c'est que nous soyons, nous souhaitons développer EDF de manière ambitieuse de manière à ce que la souveraineté économique la souveraineté électrique de la France soit assurée. Au-delà d'EDF, j'ai entendu pas mal de questions et quelques critiques. Sur le fait qu'on mettrait la charrue avant les boeufs en parlant de Saint-Arnoult et des terminaux méthaniers avant de parler de la PPE. Qu'est-ce qu'on nous aurait dit si on avait passé l'été ici et à l'Assemblée, a parlé de programmation plus réel de l'énergie à horizon des années vingt-quatre alors que la vraie inquiétude qu'on avait tous à l'époque c'est est ce qu'on aura du gaz à l'hiver, la réalité, effectivement c'est que du fait de l'invasion d'un pays souverain par la Russie. Nous nous retrouvons face à une crise énergétique que nous devons gérer et la première réponse à cette crise énergétique hé oui c'était assurer qu'on ait suffisamment de gaz en Europe suffisamment d'énergie en Europe pour répondre au risque de rationnement, que personne, je pense, sur aucun de ces bancs ne souhaite voir arriver. Alors la PPE, elle viendra, elle est prévue et elle aura une ambition, vous le savez. à la fois de développer de manière ambitieuse : le nucléaire. Et renouvelable, n'en déplaise à Monsieur Salmon, sénateur, il faut des deux sauf dans un scénario un peu extrême de RTE, nous préférons les scénarios centraux qui, de manière ambitieuse, équilibrée, ça a été dit sur tous les bancs doivent développer à la fois du nucléaire d'aujourd'hui et de demain et des énergies renouvelables à la fois de l'hydraulique, la première ministre l'a rappelé dans son intervention liminaire de l'agrivoltaïsme, vous l'avez dit aussi Madame, la première ministre en cohérence avec les voeux et les desiderata du Sénat et, pourquoi pas, la géothermie, je pense que ça a été mentionné ici également, en bref, nous sommes à l'offensive, le Sénat, le sénateur pardon, Rambaud a dit : nous sommes à l'offensive pour développer une politique énergie ambitieuse qui permettra à la France. De développer de manière durable, son industrie, j'y reviendrai en conclusion de points pour terminer : d'abord les questions qui ont été posées sur ces bancs sur le soutien au marché sur le soutien aux entreprises et sur le soutien aux collectivités locales, du fait de la crise en Ukraine et la crise énergétique qui en découlent. Beaucoup d'entre vous, certains d'entre vous ont demandé à ce qu'on supprime la reine. Oui. J'espère que vous plaisantez, le ministre de l'Industrie, que je suis, vous dit monsieur le sénateur gai que si on supprime la reine demain vous mettez toute l'industrie française à genoux à l'arrêt, aujourd'hui vous avez demandé beaucoup d'entre vous à sortir du marché européen, la réalité c'est qu'on a en partie sortie du marché européen, grâce à la reine et qu'aujourd'hui les ménages français paye une électricité qui est temps de soufre, peut-être pas le dire trop fort du tarif européen de marché et que les industriels français, aujourd'hui, s'ils sont pas tous à l'arrêt, c'est qu'une partie de leur, de l'énergie oui et payer un tarif préférentiel qui reflète l'Avantage concurrentiel d'EDF, soyons dans tous fiers et réfléchissons plutôt ensemble à la manière d'inventer le dispositif qui, au delà de la reine, puisque celle-ci sera terminée en 2023 2000 permettra à l'industrie française de continuer à profiter d'une énergie compétitive décarbonés produite par notre opérateur national. Vraiment la reine merci la reine d'abord et continuons la reine, s'il vous plaît. Demandez à tous les industriels, monsieur, monsieur le sénateur, tous les industriels m'en parle aujourd'hui, heureusement qu'on a la reine, sinon on serait mort la solidarité. Alors il va falloir changer la de la la tarification, vous avez raison, Monsieur le Sénateur Retailleau il va falloir mettre en place un découplage du gaz et l'électricité, il va falloir, on l'espère mettre en place un scénario à l'espagnole, si on l'avait mis en place au moment où vous le souhaitiez monsieur Retailleau, vous savez bien qu'on aurait subventionné toute électricité allemande et que la seule manière de faire de la solidarité nationale, madame la sénatrice hein nous l'a dit, c'est de le faire en européen et, là encore dans des polices dans déplaise aux sénateurs rêviez de le faire à l'européenne, nous gagnerons cette lutte en européen où nous la perdrons. Son soutien aux collectivités locales, monsieur le sénateur, vous avez raison de nous alerter la première ministre a déjà évoqué, nous travaillons à des situations un certain nombre à des solutions, pardon, un certain nombre ont déjà été annoncé une hausse de la dotation générale de fonctionnement de 110 millions en plus pour 2023, un filet de sécurité qui permettra d'aider les collectivités locales qui sont le plus en difficulté, bref, nous travaillons maintenant ils ne sont pas toutes en difficulté, madame la sénatrice aujourd'hui pour les industries, comme pour les collectivités territoriales, nous devons faire du ciblage un dernier point et j'en arrête là les filières industrielles, nous devons développer une énergie souveraine, nous devons produire en France ce qui va nous permettre de la produire, nous devons redévelopper des filières industrielles, ça a été dit par un certain nombre d'entre vous dans le photovoltaïque dans le nucléaire, évidemment, mais aussi dans l'éolien et pour cela, vous le savez, nous investissons, France 2030, qui fait aujourd'hui Madame la première ministre ou c'est un an, c'est exactement ça : investir dans l'innovation, de manière à ce qu'on puisse développer des filières françaises de décarbonation de l'industrie et d'industrie décarbonnées je suis extrêmement fier de participer à cette mission, qui nous permettra notamment de développer ça a été dit par certains d'entre vous, des petits réacteurs modulaires qui nous permettra, monsieur Menonville ville de fermer le cycle nucléaire de manière peut-être un peu moins dispendieux, ce que le profil Astride qui était sans doute pas très mal allez organiser et qui s'annonçait une fois de plus, comme un gouffre que nous ne souhaitons pas dépenser merci mesdames et messieurs les sénateurs, travaillons ensemble à l'avenir de la politique énergétique française, je suis sûr que nous pouvons y arriver merci. Merci, monsieur le Ministre. Pour donner la parole à Madame la première ministre. Merci monsieur le président, Mesdames et messieurs les sénateurs, en conclusion de ce débat, je veux commencer par saluer chacun des orateurs qui se sont succédés à la tribune ce soir. Les interventions ont été forte en idées plutôt qu'on polémique et chaque groupe a pu exprimer sa vision des défis devant nous. Depuis le choc pétrolier dans les années 70 régulièrement les énergies fossiles reviennent sur le devant du débat public. Systématiquement, elles sont synonymes de crise de montée des prix de menace de pénurie et de dégâts climatiques majeurs. Ce constat, nous le partageons et depuis des années, nous avançons pour trouver les moyens de sortir de notre dépendance aux énergies fossiles. Il y a quelques mois, la guerre en Ukraine, a marqué une nouvelle étape. Nous devons accélérer, je crois que c'est un consensus qui s'est dégagé ce soir un consensus que j'avais déjà observé lors des échanges que j'avais eu avec chacun des présidents de groupe. ça n'est pas la seule convergence : convergence que j'ai observé ce soir, nous sommes tous convaincus que la transition énergétique devra préserver le pouvoir d'achat des Français et conforter la compétitivité de notre économie je peux vous l'assurer, monsieur le sénateur, nous sommes déterminés à lutter contre la précarité énergétique, c'est notamment le sens du chèque énergie exceptionnel jusqu'à 200 euros pour les 40 % de Français les plus modestes, en complément du bouclier tarifaire. C'est aussi le sens monsieur le sénateur cours Corbizet de l'augmentation dans le projet de loi de finances 2023 du budget 2 MaPrimeRénov'et du maintien d'une prime à la conversion pour permettre aux Français, notamment les plus modestes, de passer un véhicule qui consomme moins. Nous nous sommes accordés aussi sur la nécessité de conquérir notre souveraineté énergétique. Nous ne pouvons plus être dépendants d'autres pays et particulièrement de ceux qui rejettent notre modèle démocratique. Nous devons être en maîtrise de notre production, c'est aussi la meilleure façon de contrôler le niveau des prix et je vous confirme, Monsieur le Président, Retailleau que nous maintiendrons le bouclier tarifaire gaz au-delà du 1er juillet avec un tarif de référence prolongé pour les années suivantes, je vous confirme également que nous travaillons depuis des semaines pour mettre en oeuvre ce modèle ibérique à l'échelle européenne car, contrairement à l'Espagne, nous ne sommes pas une péninsule nous sommes fortement interconnectés avec les autres États membres la nécessité, c'est d'avancer à l'échelle européenne. Et par ailleurs, Monsieur le Sénateur, Gay, je vous confirme que nous voulons aussi une réforme durable du marché de l'électricité avec un découplage des prix du gaz et de l'électricité je je suis et je reste convaincu que notre souveraineté passe par la France et par l'Europe. Ce soir, bien sûr, j'ai aussi entendu quelques caricatures ou procès d'intention. n'est pas forcément utile de polémiquer car nous savons aussi que ça n'est pas sur une année ou même sur quelques années que se jouent les transformations dans la filière nucléaire, elle se joue sur des dizaines d'années ce qui, bien avant nous, ont lancé le programme nucléaire français, le savait parfaitement. Personne ne l'ignore, ici il y a eu au cours des 25 dernières années pratiquement tous les 5 ans des alternances politiques. Au cours de ce chemin, peut-être y a-t-il eu des erreurs et si c'est le cas, je pense à tout le moins, quelles sont partagés. Et si nous devons être lucide, il faut l'être jusqu'au bout, la France a fait le choix de préserver son parc nucléaire, il dit : investir. Certains de nos grands voisins n'ont pas fait ce choix et nous pouvons être fiers de la confiance que nous avons toujours placé dans notre filière nucléaire confiance aussi dans notre grande entreprise nationale EDF qui ne saurait être question de démanteler. Au cours de nos débats, c'est au tour de notre mix énergétique que j'ai entendu la plus forte différence d'approche, je l'ai dit, je l'ai dit tout à l'heure et je le répète devant vous, ma conviction est qu'un mix diversifié nous protège et garantit notre souveraineté. Car il n'existe pas d'énergie sans défaut. Je le disais, nous croyons fermement au nucléaire, nous sommes convaincus qu'il s'agit de la voix de l'efficacité de la souveraineté et de la neutralité carbone. Mais nous ne pouvons pas non plus faire croire que c'est une énergie tout à fait banal. Merci. Le le chantage russe autour de la centrale de Zaporijia nous le rappelle durement, nous ne pouvons pas nous permettre non plus de tout miser sur une seule source d'énergie en cas d'avarie de problèmes techniques ou de défaut, nous serions alors exposé démunis, nous voulons donc développer aussi sans hésiter les énergies renouvelables. Elles sont décarbonés bénéfiques pour notre économie, elles permettent l'émergence de nouvelles filières industrielles et ses apports énergétiques sont déterminants, particulièrement dans les moments de tension cependant nous n'oublions pas qu'elles sont intermittentes et pose des questions d'acceptabilité, elles ne peuvent pas être seule l'Alpha et l'oméga de notre action énergétique, même si, comme vous l'avez souligné madame la sénatrice, Denise Saint-Pé, elles peuvent aussi constituer un complément de revenus pour nos agriculteurs, qu'il s'agisse de l'agrivoltaïsme ou de la méthanisation je crois donc à l'équilibre à la diversification et avec mon gouvernement, nous continuerons à les défendre. Mesdames et messieurs les sénateurs, les échanges de ce soir, ouvre une séquence nous posons d'abord les termes de notre débat, nous aurons ensuite à discuter dans les prochaines semaines de de projet de loi d'urgence pour accélérer le développement de nos énergies renouvelables et nos projets nucléaires enfin une fois les débats sous l'égide de la CNDP qui démarre actuellement menée, nous pourrons débattre en 2023 d'une loi de programmation énergie climat je souhaite et j'espère que l'esprit de responsabilité et la volonté d'agir, dont nous avons fait preuve ce soir nous guideront collectivement dans les échanges à venir, vous pouvez compter sur moi et mon gouvernement pour écouter chacun et chercher des compromis sur l'énergie, en particulier, je suis convaincu qu'ils sont à notre portée, je vous remercie. Mes chers collègues, je vais maintenant lever la séance, notre prochaine séance aura lieu demain jeudi 13 octobre à 10 heures 30 pour la suite du projet de loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur, la séance est levée.